La séance est ouverte, le compte rendu analytique de la précédant l'séance a été distribué, il n'y a pas d'observation, le procès verbal est adoptée sous les réserves d'usage. Par lettre en date du mercredi 15 novembre 2017 Monsieur monsieur Jean Bizet, président de la commission des affaires européennes a demandé l'inscription alors du jour d'un débat préalable au conseil européen des 14 et 15 décembre 2017 ce débat pourrait être inscrit alors du jour du mardi 12 décembre 2017, à l'issue du scrutin public à la tribune sur l'ensemble du projet de loi de finances pour 2018 il y a-t-il des observations. Il en est ainsi décidé. Lors du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'amendement 14 rectifier qu'inquiet tendant à insérer un article additionnel après l'article 35. Monsieur Deriot vous avez la parole pour eux, cet amendement. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mais chers collègues oui ce cet amendement concerne le dossier pharmaceutique qui est un dossier électronique partagé contenant les informations sur les médicaments dispensés aux patients au cours des 4 derniers mois dans l'ensemble des pharmacies françaises en ville comme à l'hôpital, cet outil permet aux pharmaciens de détecter d'éventuels surdosage ou contre-indications ces informations seraient également utile au pharmacien biologiste, car les traitements pris par les patients peuvent influencer les résultats des examens de biologie médicale et impacté l'expertise du biologiste

le biologiste doit, en effet, le cas échéant alerter le patient et le prescripteur afin que ce dernier a juste de la prescription de plus, la connaissance des médicaments pris par les patients est indispensable car certains médicaments interfère avec les méthodes de dosage en biologie médicale, par exemple, c'est le cas de la Bugatti qui a fait l'objet d'ailleurs d'une alerte récente de l'ANSM par ailleurs, l'ensemble des médecins, des établissements de santé ont aujourd'hui accès au au dossier pharmaceutique les médecins biologistes donc des établissements de santé ont donc accès à ces données, à l'inverse des pharmaciens biologistes de ces établissements, c'est pourquoi il serait nécessaire qu'il puisse également être je rappelle que les pharmaciens biologistes représentent 80 pourcent des biologistes en France qui me paraît quand même indispensable, je vous remercie. Merci l'avis de la commission madame. La, la Commission a jugé cette évolution en effet tout à fait pertinent, même si on peut s'interroger, savoir c'était la place dans un PLFSS mais elle est en effet susceptible de contribuer à la paieront finance et à la qualité des soins et elle a mis un avis favorable. Mohamed madame la milice favorable aussi, il y a-t-il des explications de vote. Il y en a pas, qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Cet amendement est adopté, nous passons à après l'article 35 l'amendement 96 rectifier Madame Cohen monsieur votera oui merci. Nous avons bien lu le plan présenté par le gouvernement pour renforcer l'axe et territoriale, aux soins, il prévoit de lutter contre les déserts médicaux en fournissant des aides supplémentaires l'installation facilitant le cumul emploi-retraite des médecins libéraux ou les pratiques mixtes, par exemple, mais je peux bien évidemment pas tout citer si ces mesures ne semble pas différer fondamentalement dans leur philosophie des incitations mises en place par les gouvernements précédents qui ont fait la preuve de leur échec, malheureusement, je sais qu'il y aura une évaluation, c'est un progrès cependant les données statistiques disponibles semblent confirmer l'analyse du géographe de santé Emmanuel Vigneron, qui conclut que, sous l'effet de la métropolisation, je cite, les fractures se sont agrandies et de vastes pans du territoire sont désormais en voie de désertification, je prendrai l'exemple de mon département, le Pas-de-Calais, à la fois très rural et très urbain ou il ment globalement 200 généralistes et plus de 1000 spécialistes pour atteindre la densité moyenne nationale alors que le taux de surmortalité évitable, les taux de surmortalité évitable bat tous les records, si dans la métropole lillois, celle-ci est largement supérieur à la moyenne du fait de l'attractivité du CHRU, c'est le contraire dans certains territoires du Pas-de-Calais département injustement privé de CHU dans le sein peut loi très rural, la densité médicale atteint péniblement la moitié de la moyenne nationale, dans le bassin minier, particulièrement touchée par les problèmes respiratoires dont a parlé le ministre Darmanin du fait de son histoire, le service de pneumologie de l'hôpital de Lens vient de fermer, de même que celui de cardiologie de l'hôpital de Béthune, faute de spécialistes à Auchel, dans le centre de santé quinze spé telle spécialité, celui-ci vient de fermer et les moyens obtenus de la RS grâce à l'action des élus pour mener le dépistage Ratinho diabétiques et réinstallé 2 fauteuils dentaires ces moyens ont dû être abandonnés car aucun ophtalmo aucun chirurgien dentiste n'a voulu venir sur ce territoire de l'ouest du bassin minier particulièrement frappés par la crise, alors il ne s'agit pas pour nous d'instruire un quelconque procès contre les médecins mais de faire le constat de l'insuffisance, voire de l'échec des mesures incitatrice déjà prise au regard de de la désertification médicale et de l'impératif d'égalité des citoyens devant la maladie, tels le sens de notre amendement qui, à l'image de ce qui est demandé aux jeunes enseignants demandent aux médecins désireux d'exercer leurs fonctions à titre libéral de s'installer pour une durée d'au moins 2 ans dans un territoire sous-dotées. Alors, cet amendement est le 1er d'une série puisqu'on va aborder la question de la liberté d'installation des médecins. Au regard des enjeux-là, que ce soit dans notre territoire je m'exprimerai un peu plus longuement sur ce gel sur les amendements qui suivent, mais la commission est défavorable à cet amendement qui recourt à la contrainte pour l'affectation de je ne tiens la sortie de leurs études, cela ne serait pas de nature à renforcer l'attractivité de l'exercice libéral une une position que la Commission défend depuis depuis longtemps. Madame la ministre. Oui, Monsieur le Président, comme vous le savez nous venons présenter un plan d'accès territoriale aux soins, nous avons souhaité changer de paradigme et ne pas tout miser sur l'installation des médecins dans des territoires qui, de fait, manque d'attractivité pour X raisons et et je ne reviens pas là dessus parce que cette politique colère atteint ses limites quand il s'agit d'une profession dont la démographie est faible, c'était une procédure qui est utile, par exemple, qui a été utile pour réguler l'installation des infirmières qui était une profession surdotées mais lorsque l'on manque de médecins dans tous les territoires, les politiques merci tive vont favoriser le fait par exemple que les jeunes femmes médecins qui sortent de la faculté n'iront pas en zones sous-dotées de façon sommaire mais préférant prendre un un travail salarié éventuellement comme médecin du travail au médecin scolaire où il en manque, par dizaines, et donc je pense que nous n'entendons pas notre but, c'est la raison pour laquelle, dans le plan d'accès territoriale aux soins plutôt que de tout miser sur l'installation, même s'il y a des mesures incitatives qui persistent pour l'installation, nous avons proposé qu'il y avait du temps médical projetés dans les séries Touaregs sous-dotées, donc nous misons plutôt pour une réorganisation de l'offre de soins des du temps médical est donné soit par un hôpital de proximité, soit par les médecins libéraux du territoire avec une forme de responsabilité territoriale qui est donnée au c'est et aux hôpitaux sous avec la RS, qui doit se mettre en ordre de marche pour organiser le territoire de cette façon-là avec beaucoup de mesures incitatives à ce que des médecins a et donné du temps médical, notamment avec une revalorisation du C de la consultation de 25 pourcent avec des postes partagés d'assistants entre les hôpitaux et des zones sous-dotées en favorisant la découverte avec de l'exercice libéral auprès des jeunes, que ce soit des externes et des internes en zones sous-dotées et donc beaucoup de mesures incitatives dans ce sens, par ailleurs, il existe déjà des contrats de service public qui sont qui qui ont pour vocation à faire en sorte que des jeunes médecins s'engagent à aller en zones sous-dotées, si on leur donne une bourse d'études, une une démarche la volontaire 1795 contrats de ce type ont été signés à ce jour et cela, vocation à perdurer, donc je suis défavorable à votre amendement, même si, bien entendu, nous partageons le constat de la difficulté sur le territoire. Bien je vois qu'il y a des demandes d'explications de vote Madame Goulet. Monsieur le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues, j'ai bien entendu ce qu'a dit le ministre, et c'est vrai qu'on qu'on attend un plan intelligent qui qui laissent faire les les territoires et qui permettent les expérimentations, c'est ce que vous avez Madame proposé évidemment on est, on est tout à fait favorables à cela, néanmoins je vais par principe soutenir, ne serait-ce que pour pour le principe, c'est l'amendement déposé par nos collègues et les mesures de contrainte, je sais qu'elles ne sont pas efficaces mais je sais que, en même temps on les a jamais vraiment essayer, on les avait voté dans la loi Bachelot hôpital, patients, santé, territoires, elles ont été votées au Sénat, elles ont été votées à l'Assemblée nationale, puis une proposition de loi UMP à l'époque, est revenu sur la disposition qui avait été voté dans le texte hôpital, patients, santé, territoires, c'était une mesure de bon sens. Et moi, par principe, je je voterai donc l'amendement proposé par nos collègues. Le président Millon a demandé la parole, mais il y a encore 3 interventions préféré après ou tout de suite. Après, très bien monsieur Amiel. Oui, le mode d'exercice tels que ben, entre autres, je l'ai pratiqué pendant 35 ans, est désormais terminée, la démographie médicale est très défavorable, et cela va s'aggraver, d'après les les chiffres jusqu'en 2025, alors ma crainte concernant les mesures courir City veut c'est que cela aggrave encore les choses, pourquoi le choix de faire de la médecine, il faut 10 ans pour faire un match, ce sont des études longues, ce sont qui a, qui annonce un métier plutôt difficile, si on dit encore à des jeunes gens qui veulent qui veulent prendre les études médicales, à la fin, ils vont se retrouver face à des mesures Commercy TIW j'ai peur que on les décourage encore bien davantage, on a évoqué je l'évoque moi-même ici la question du numerus clausus, comme si c'était une panacée de dire ouvrant largement le numerus clausus, quand on sait comment se passent les études médicales dans l'université, que l'hôpital ne peut pas accueillir massivement, je dis bien massivement de, d'étudiants, mais de ceux qui le font, ils le peuvent, anti-peu mais de façon finalement assez marginal, alors l'intérêt de ce qui est présenté là c'est effectivement comme vous l'avez dit Madame la ministre, nouveau paradis l'utilisation de la télémédecine, le décloisonnement ville hôpital dans les Bouches-du-Rhône, où il y a des disert médicaux, contrairement à ce qu'on peut imaginer, on a fait quelques ici où les praticiens libéraux et hospitaliers viennent travailler ensembles incontestablement le mode de changement de rémunération le les rémunérations paiement à l'acte, beaucoup de jeunes médecins n'y sont plus attachés, ils veulent vivre normalement aux c'est-à-dire finir leur journée à des heures normales, ne pas être appelé la nuit ne plus prendre des gardes et je mets pas forcément en avant la féminisation de la profession, c'est un changement sociologique, c'est, c'est c'est c'est quelque chose de de tout à fait normal, donc j'ai envie de dire, bon, on fait là des propositions qui sont quand même novatrice évaluons les d'ici 3 ans parce que je pense qu'on ne peut pas pour un schéma comme celui-là, dira bah on verra dans 6 mois, ce qui se passe, puis dans 3 ans, peut-être qu'il faudra re revoir ces mesures prises mais à l'heure actuelle, je suis très défavorable aux mesures Quincy. Merci Madame Cohen. Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, je trouve que les mesures incitatives qui ont été énoncés par Madame, la Mini sont. Intéressante mais je pense que les remèdes face aux déserts médicaux sont vraiment multifactoriel et que ce débat est primordial dans notre dans parce que, effectivement, notre collègue vient d'. Parler du numerus clausus nous au groupe communiste, républicain, citoyen écologiste, on est pour sa suppression continue de la gravité de la situation aujourd'hui est contenu du fait que il faut 10 ans pour former des médecins. Vous parlez de décloisonnement entre la ville et l'hôpital bah moi vraiment je suis franchement d'accord j'ai faut qu'on arrête d'opposer les pratiques médicales, donc tout à fait d'accord, mais en même temps, Madame la Ministre,

mais on a fait avec mon collègue Dominique Vatrin travail autour de nos 3 départements avec Annie David, qui était présente dans cet hémicycle, Isère, Pas-de-Calais et Val-de-Marne on a rencontré des des professeurs de de médecine qui travaille en milieu hospitalier, on a rencontré des proches libéraux, quand on a testé cette mesure qui apparaît, une mesure de vraies vraiment colère City, ils ont, il y a pas eu de tollé comme il pouvait y avoir quelques années en arrière, parce que tout le monde est conscient de la gravité de la situation, donc je pense qu'il faut réfléchir, y compris à ces mesures-là, évidemment, là où je suis d'accord c'est que ça va, c'est un tout, c'est-à-dire qu'un un médecin ne va pas aller s'installer, même pour 2 ans dans un endroit où par exemple il n'y a pas de service public, il n'y a pas d'école etc

Merci Monsieur le Président, je voulais pas intervenir sur tout ce qui a été dit par Madame la ministre par Madame rapporteur ou même par Michel Amiel, puisque je suis complètement d'accord avec tout ça, moi je voulais intervenir sur le fait que régulièrement on entend dire que les étudiants en médecine coûte cher, je dirais que, a priori, j'ai sentiments que tous les étudiants dans toutes les disciplines, coûte cher à ce moment-là les étudiants lettres également étudiant en droit également etc faut arrêter d'essayer comme ça de, de, de stigmatiser des étudiants plutôt que d'autres, les étudiants en médecine, en plus, coûte certainement moins cher que beaucoup d'autres, puisque dans leurs études de médecine, ils doivent aller dans les hôpitaux, il travaille dans les hôpitaux et dans les hôpitaux ne sont pas rémunérés, donc il ne coûte, c'est probablement moins cher que beaucoup d'autres, ils font un travail qui n'est pas faite évidemment par des salariés et au bout du compte, si on fait le calcul de l'ensemble ne coûte pas si cher que ça, c'est le 1er point le 2ème point lorsqu'ils sont devenus médecins et pour devenir médecin, il faut qu'ils soient évidemment encadré par des professeurs de médecine par des chirurgiens par des médecins par des praticiens hospitaliers, il faut donc qu'ils soient en contact Direct avec le patient avec leur patron avec leur patron avec ceux qui savent, avec leur sachant et cela ne peut se faire que s'ils sont en nombre suffisant mais pas en surnombre, si jamais vous libérer numerus que ZUS, vous allez voir un surnombre d'étudiants obligatoirement qui n'auront pas le contact avec les sachants et qui est vous ferait à ce moment là des des médecins qui n'auront pas la connaissance suffisante pour être efficace dans dans leur métier, enfin, pour terminer la coercition n'a jamais chez je parce que dire : souvenez-vous de la prohibition. Merci, il n'y a plus d'explications de vote, je vais vous consulter

voir en allant si c'est efficace ou pas, donc ça là dessus, on est OK, vous avez dit que dans le contexte d'une démographie médicale très faible si on impose une contrainte, il aura un effet pervers et une fuite vers le salariat, moi je trouve pas que c'est un problème, au contraire, moi je pense que d'ailleurs, quand on est, on propose des directif Eschauer City fallait n'hésitons pas d'utiliser le mot ça vaut pour la mesure clé dans cet amendement, ça vaut aussi pour l'État pour la sécurité sociale qui doivent investir sur ces territoires pour faciliter l'installation de Centre de santé par exemple, parce que globalement il y a une majorité de jeunes médecins des d'étudiants en médecine qui sont pas contre l'exercice salarié de la de la médecine sur le numerus clausus, nous on a toujours été dans notre groupe, contre la mise en application, on en paye les effets, on voulait faire des économies à l'époque, hé bien aujourd'hui on paye les effets mais on a beau augmenter le nombre de places dans le cadre des CHU quand il y a pas de CHU dans un département du Pas-de-Calais d'un 1000000 500000 habitants n'a pas les effets j'ai vu que vous aviez lancé Madame la ministre, une mission pour un CHU moderne dans laquelle il y aura cette objectif de, de, de combattre les inégalités territoriales, je, je, je m'inscris pleinement dans ce dans cette démarche et je vous demanderai bien évidemment un rendez-vous avec les élus de mon territoire. Merci de nouvelles inscriptions dans le débat Monsieur Touraine. Je justement où je suis un peu

Quant par les professeurs et qu'on on on exige de un certain nombre de contraintes, on n'a pas les mêmes réactions et je pourrais évoquer l'ensemble des des professions pas dire pour autant qu'il faille le faire mais tout de même, il n'est pas interdit d'en discuter et ça n'est pas faire affront à cette corporation dont on a tellement besoin de la même façon, dire que les études de médecine coûtant ça n'est pas les stigmatiser CDC objectif et, par conséquent, moi je, alors on peut effectivement discuter intégrer peut-être un certain nombre de services non rémunérés qui sont, qui sont offerts le dessus, je suis un peu étonné de de certaines réactions. Merci Monsieur

mais il faut savoir quand même que les les élus sont absolument désespérée parce que sans médecin dans un territoire ça va entraîner, c'est la première désertification qui va arriver, alors j'espère, et justement je je ne voterai pas, même si je suis d'accord sur le sur le fond avec ce cet amendement, je ne voterai pas parce que j'espère que les solutions nouvelles que propose Madame le Ministre, qui a été dit l'emploi salariés une possibilité d'être salarié de nouvelles de nouvelles initiatives permettront de trouver une solution j'ajouterai quand même que le numerus clausus pour moi doit être augmentée, et je pense que il faudrait un internat par faculté, avec aussi des idées, des stages et bien sûr des maîtres de stage qui soient peut-être mieux considérés, mieux rémunérés, mais un internat par faculté et un stage de 6 mois chez le praticien comme à l'hôpital, merci. Merci madame le rap, oui. Rapidement, c'était pour répondre à Monsieur Touraine, en nous disant le professeur oui, sauf que les professeurs se sont des fonctionnaires, alors on peut avoir le débat, on peut avoir le débat, mais à ce moment-là on dit voilà les les médecins seront fonctionnaires, ils seront en toute connaissance de cause lorsqu'ils commenceront leurs études, mais allez dire à des étudiants sur des études qui dure 10 ans, voilà, il y avait une projection de l'exercice de profession que celle-ci est maintenant, hé bien non, vous installeraient là on voté vous installer, je trouve que ce n'est pas raisonnable 2 ans 2 ans oui c'est ça après 10 ans d'études. Et nous passons au vote qui est pour. Qui compte. Qui s'abstient cet amendement n'est pas adopté alors après l'article 35 il y a six amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Madame Meunier, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président Madame réalisme cher collègue, nous sommes dans le même sujet et donc là peut-être qu'il y a un peu moins de coercition, un peu plus d'incitation, mais c'est le même objet, donc le constat il est partagé par chacun et chacune d'entre nous ici ne faisons rien, c'est déjà trop tard, ce sont bien sûr la Les petites communes les moyennes communes mais aussi tout le secteur périurbain et parfois le coeur des villes qui est concerné par ces difficultés d'installation donc cet amendement, il a pour but de lutter contre l'aggravation du phénomène et et il est temps aux médecins libéraux, un dispositif de régulation à l'installation, qui existe déjà dans d'autres domaines de professionnels de santé, les infirmières, les masseurs kinésithérapeutes, les sages-femmes, etc donc, il prévoit l'amendement que dans des zones définies avec les ARS et en concertation avec les syndicats médicaux, un nouveau médecin libéral ne peut s'installer en étant conventionnés à l'assurance maladie que lorsqu'un médecin libéral de la même zone cesse son activité, le principe de la liberté d'installation demeure donc, mais le conventionnement n'est possible que de manière sélective pour ces nouvelles installations voilà je merci. Merci. Alors, le 310, là on est sur 4 amendements identiques, donc les balaye tous 310 rectifier sexy, il n'y a aucun présent des signataires, donc il n'est pas défendu ils tombe me scientistes pour le 421 à rectifier bis. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Michel collègues les derniers chiffres publiés le 12 octobre 2017 par l'Ordre des médecins concernant la démographie médicale sont particulièrement alarmants presque partout en France, notamment pour la médecine générale à situation est également inquiétante pour certaines spécialités médicales. Dans le but de lutter contre l'aggravation de ce phénomène, le présent amendement étend aux médecins libéraux, un dispositif de régulation à l'installation, qui existe déjà pour plusieurs autres professionnels de santé, pharmacies, infirmiers masse qui n'hésitez sage-femme chirurgiens dentistes, orthophonistes, il prévoit que dans des zones définies par les ARS en concertation avec les syndicats médicaux dans lesquelles existe un fort excédent en matière d'offre de soins un nouveau médecin libéral ne peut s'installer en étant conventionnés à l'assurance maladie que lorsqu'un médecin libéral de la même zone ça son activité, le principe de la liberté d'installation demeure donc, mais leur conventionnement n'est possible que de manière sélective pour les nouvelles installations, l'adoption d'une telle principe de conventionnement sélectif des médecins libéraux permettrait de compléter utilement le dispositif d'incitation à l'installation dans les zones sous-dotées, qui ont été mises en place dans le cadre du pacte et 3 en matière de lutte contre les déserts médicaux, il est en effet urgent de mobiliser l'ensemble des solutions possibles, en particulier lorsque celles-ci ont déjà fait preuve ont déjà fait leurs preuves pour d'autres professions de santé, merci.

Monsieur le président, la ministre un amendement effectivement qui va dans le même sens, la désertification médicale connaît actuellement dégradation inquiétante, on vient d'en parler, la Cour des comptes dans son rapport annuel sur l'application des lois de finances de la Sécurité sociale présente en septembre 2007 partage ce constat le ce constat, écrit la concentration géographique tend à s'accroître et les écarts de densité médicale sont considérables des départements entiers sont désertés par certains spécialistes, elle préconise l'instauration d'un conventionnement sélectif des spécialistes est amendement propose la mise en oeuvre de cette recommandation. ah non non on oui, oui, on a fini avec les identique. Nous poursuivons avec les amendements de la discussion commune toujours madame Meunier, pour le 208. Rectifier 1er. Oui, donc c'est un peu près la même chose sauf que comme on veut être source de propositions presque un amendement de repli, parce que, à cette recommandation numéro un caractère expérimental, pour une durée de 3 ans est assorti d'une évaluation au bout de 6 mois, un an pour évaluer tout le bénéfice de cette incitation à l'installation des médecins libéraux.

Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, l'amendement que je présente prévoit une expérimentation, le mot est important, le conventionnement collectif que cette expérimentation puisse être menée sur une période de 3 ans dans les zones dites surdotées, c'est-à-dire les zones dans lesquelles existe un fort excédent en matière d'offre de soins, la fracture sanitaire ne cesse de s'aggraver et les politiques incitatives mises en place depuis 25 ans ont montré leurs limites, les mesures proposées récemment par le gouvernement pour lutter contre les déserts médicaux continuons dans cette voie, ne prennent pas toute la mesure du problème qui touche le territoire, il semble donc nécessaire d'aller au-delà aussi cet amendement propose que dans les autres zones dites surdotées définie par les ARS en concertation avec les organisations représentatives des médecins, un nouveau médecin libéral ne puisse installer en étant conventionnés à l'assurance maladie que lorsqu'un médecin libéral de la même zone cesse son activité. Le principe de la liberté d'installation demeure mais le conventionnement n'est possible que de manière sélective pour les nouvelles installations, ce système de régulation reposant sur le conventionnement sélectif existe déjà pour la plupart des professionnels de santé, les infirmiers, les sages-femmes, les orthophonistes échange un dentiste et a largement fait ses preuves dans ses différentes professions en choisissant le principe de l'expérimentation, c'est amendement permettra d'évaluer sa pertinence avant d'envisager sa pérennisation pour ce faire, 6 mois avant la fin de l'expérimentation, cet amendement prévoit que le gouvernement remette un rapport au Parlement afin d'évaluer son impact merci. Merci donc la vie madame la rapporteure, l'avis de la Commission sur cette. Oui, j'ai donné un avis global, hein, puisque c'est un avis défavorable sur l'ensemble des amendements, que ce soit sur le conventionnement sélectif avec le conventionnement uniquement en cas de remplacement d'un d'un médecin partant à la retraite ou sur l'expérimentation lors de précédents débats et avait été notamment le cas lors de l'ordonnance Santé, la commission s'est opposée à l'instauration de ce dispositif d'un conventionnement sélectif qui rejetée par médical mais notamment par les internes et les jeunes médecins et à la suite de de ces débats, souhaite la loi santé soit du nez précédent PLFSS la la AM-EX ça conduit au 1er semestre une mission sur les dispositifs incitatifs en faveur de l'offre de soins dans les zones sous-dotées, alors le rapport nos collègues Jean-Noël Cardoux Yves Daudigny qui a été publié en juillet dernier, avance de nombreuses propositions pour agir au plus vite et et plus efficacement mais confirme la position de la Commission, un sujet sans négociations avec les professionnels de santé concernés sans leur assentiment une évolution de cette nature pourrait être inefficace au regard des enjeux des zones sous-dotées, en effet, ce dispositif pourrait détourner des jeunes médecins d'exercice en libéral, voire de l'exercice, la médecine tout court et en août l'instauration du du principe une installation pour un départ dans les zones surdotées n'apportent nullement la garantie d'un rééquilibrage géographique. De l'offre de soins au profit des zones sous-dotées, le conventionnement sélectif a été mis en place, mais avec l'accord de la profession pour des infirmiers dans un contexte démographique très différent de celui des médecins, on avait une sur un surnombre de de professionnels, ce qui est pas du tout le cas pour les médecins, or on constate des effets de contournement avec des installations à la lisière des zones, des zones dites sur Danse et un à pacte finalement assez limité sur les zones les plus fragiles en termes d'accès aux soins, cela est également constatée lors de la mise en place de cette mesure en Allemagne, comme l'avait souligné un rapport, publié l'an dernier par la note rapporteur général et par Yves Daudigny, alors bien sûr ce ce cette notion d'accès aux soins, les cruciale on l'entend sur sur tous les bancs de l'hémicycle, on l'a vu, ça suscite à la fois des inquiétudes forte des élus et et nous par exemple en région Pays de la Loire, lorsqu'on a fait une enquête sur la ruralité, c'est avec l'accès au numérique, la 2ème préoccupation des élus, c'était celui de l'accès aux soins, même si les problèmes de de démographie médicale et et d'installation, il ne touche pas que les zones rurales, on a des zones rurales qui se sont organisés : c'est le cas du département de la Mayenne en territoire très très rural, Madame la Ministre, c'était d'ailleurs où il y a un pôle santé en milieu hyper râle mais qui qui fonctionne remarquablement bien parce qu'il y a eu une prise, une prise en en compte de la situation des de l'ensemble des professionnels de santé, médicaux ou paramédicaux et et qui se sont organisés au vrai autour d'un vrai projet de santé de territoire, donc ça n'est pas que rural, ça peut être pire urbain et ça peut être des quartiers d'huile et ce n'est pas qu'une question de médecine libérale une médecine salariée on actuellement, un centre de santé au Mans qui n'arrive pas à réellement c'est quand même pas une ville totalement paumé en pleine campagne et c'est plutôt près de Paris, et qui n'arrivent pas à trouver de médecin salarié donc le le problème est beaucoup plus complexe que ça, il y a pas de solution miracle, c'est vrai, mais je pense que dans le plan que qu'a décliné, madame la ministre, dans ça sa stratégie d'accès aux soins, c'est la la multitude de mesures qui vont pouvoir qui vont pouvoir aider à résoudre, je pense que il y a à la fois bien sûr le développement des maisons de santé pluri-professionnelle ou des centres de santé ainsi dans dans certains secteurs, l'exercice de la médecine salariée et celui qui ont conduit au territoire il y a aussi, et quand je dis maisons de santé, ce sont pas des murs, hein, on voit beaucoup d'élus qui construisent des coquilles vides, en se disant je vais construire des dépôts, centres de santé et et ils viendront, mais non, c'est l'exercice coordonné et ses projets de santé du territoire de tous les professionnels, donc il y a ça, il y a aussi le développement, en effet, des stages en dans les maisons de santé qui donne aux étudiants le goût de de l'exercice libéral, il y a aussi lors des formations, faire en sorte que les professionnels de santé, toutes tendances confondues, que ce soit les les IFSI ou dans un centre de formation que dès le départ, on arrive à les faire travailler ensemble pour qui qui soit préparés à l'exercice pleurer professionnel il y a les maisons de santé, les professionnels, universitaires et son développement en Pays de la Loire et de la région va soutenir une expérimentation la la faculté de Nantes ou ou des projets de recherche en soins primaires vont être exercée dans l'Les des maisons de santé multiples où il y aura la faculté et le CHUV vient au contact de du territoire, donc je pense que c'est la conjonction de toutes ces mesures qui peuvent faire que que des jeunes médecins à l'issue de de leurs études, parce que sur 100 qui sortent, il y en a 25 qui ne sont pas inscrits à l'ordre donc déjà ont disparu des radars, si je puis dire, donc il faut les inciter très tôt et leur leur montrer ce que l'exercice de cette profession, mais ça passe aussi par le partage des tâches et des actes soit fait ce qu'il faut, c'est que les médecins puissent exercer dans des conditions qui sont celles qu'ils attendent que le territoire soit suffisamment accueillant aussi pour le travail du conjoint pour il faut qu'ils puissent exercice en exercice multiprofessionnelle, les médecins ont un peu peur, d'exercer seul donc c'est toute toute une dynamique tout à fait nouvelle qu'il faut créer près de l'offre de soins et l'article 35 à cet égard, va, va nous aider, mais je pense que des mesures comme ça qui paraît séduisante, en effet, on a tous un moment de dire, mais il y a pas de médecins obligé à venir si on est territoire c'est ce que nous disent les maires dans nos départements, je pense que ce sera contre-productif et puis les histoires de zonage,

et puis, et puis surtout un détournement d'un exercice libéral, on a déjà, il faut déjà incité les jeunes à faire c'est exercice de médecine généraliste parce que souvent auprès d'études très longues, parfois, ils ont tendance à aller vers la spécialité plutôt que de la médecine générale, mais je pense que les mesures telles qu'elles sont définies serait contreproductif et c'est finalement une

Quand vous demandez la parole, vous l'avez quand vous voulez donc où vous c'était pour compléter. Vous me dites. Ravachol, donc on on a le temps, madame la Ministre votre avis sur cette série. Oui, monsieur le président, Mesdames rapportera a tout dit mais moi j'ai une question à vous poser, parce que vous représentez les territoires, la Chambre haute, je voudrais savoir lequel d'entre vous considèrent qu'il est dans une zone sous surdotées en médecins. Qui lève la main et les 10 ans qui viennent vont s'aggraver, donc nous avons tous sans tête, une ou 2 villes peut-être pourrait considérer qu'un trop plein de médecins mais par exemple Paris, nous savons que Paris n'est pas une zone sur-dotée aujourd'hui vous attendez 6 mois pour avoir un rendez-vous d'ophtalmo, donc c'est une fausse bonne idée, il n'y a pas de zones surdotées donc on connaît les phénomènes de contournement Madame Desroches les a dit vous êtes bien placé pour savoir dans les territoires, la densité de médecins, je ne pense qu'il n'y a pas un seul entrevue aujourd'hui qui considère qu'il est dans une zone surdotées quand on voit les difficultés du zonage pour les zones sous-dotées, je ne vous parle pas de la difficulté du zonage pour les zones surdotées, donc c'est une fausse bonne idée et donc je suis défavorable bien entendu. Bien, merci, il y a des explications de vote Monsieur Savary. Oui merci effectivement moi je partage tout à fait l'avis de de Madame la la ministre offert attention parce que si on veut encourager les étudiants à aller dans la médecine générale, faut pas leur donner des si négatif parce que sinon ils vont aussitôt choisir une autre filière. On y a tous pensé, ça pouvait être effectivement une idée parce qu'on est tout cela va faire un constat on voudrait on voudrait en milieu rural ayant exercé en médecine de groupes, je peux vous dire que quand on a proposé aussi un certain nombre de choses, on arrive finalement à à faire en sorte que les jeunes reviennent, moi j'ai l'impression que les choses s'améliorent et elles s'améliorent encore si on donne plus de souplesse, donc les propositions qui sont faites à travers le plan santé me paraissent tout à fait innovante pour leur donner un petit peu d'chance notamment hier j'avais réagi par rapport au au au remplaçant un médecin généraliste en fait en ambulatoire ou nomade, mais finalement, pourquoi pas, pourquoi pas, parce que effectivement il pourrait y avoir une approche complètement différente, on sait que le médecin de famille, telle qu'on l'a exercée pour un certain nombre de qui était médecine extraordinaire n'existera plus, mais si on veut contraindre les personnes s'installent et ça veut dire qu'il faut les prévenir quand elles font leurs études, donc c'est au départ, c'est aujourd'hui pour dans 10 ans, à ce moment-là, autant ouvrir un peu plus ce numerus clausus en réglera le problème, hein, parce que s'il y a 10 ans, on avait, on fait tous le constat qui n'a pas assez de médecins. Bon, s'il y a 10 ans, on avait ouvert un peu plus, aujourd'hui, on ne serait pas où il y a 15 ans, on serait pas face à ces difficultés, donc moi ce que je crains quand même c'est que il faut un peu plus de médecins, même s'il y en a jamais eu autant parce que c'est l'évolution des choses avec le vieillissement etc de la population, donc on n'échappera pas, il y a, à ce moment-là il y aura une liberté complète, il y a plein médecin qui en véritablement travail à qui les patients font confiance, qui vont trouver à s'installer quand on forme des ingénieurs ou ou d'autres formations scientifiques ou littéraires avec des poches de doctorants post-doctorants, ça on les oblige pas s'installer, il y a peut-être moins de missions de service public, mais il n'empêche que l'attractivité me paraît plus importante pour fournir des personnes dans une profession que la coercition, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il vaudrait mieux retirer cet amendement, mes chers collègues. Mouillé. Oui, merci Monsieur le Président, juge pour faute profite pardon de de cette discussion pour vous faire part d'un témoignage, puisque dans ma commune, en tant qu'élu dans une zone un peu compliqué, j'ai l'occasion de travailler sur la mise en place d'une santé avec la venue de 4 jeunes médecins et au-delà de tout ce qui a été évoqué dans par la banale, rapporteur sur le le projet de santé sur la mutualisation, moi je voudrais vraiment insister sur 2 faits marquants en tant qu'élu local, je suis pas médecin mec sur lequel j'ai été très fortement impliqué, d'abord c'est la relation avec l'hôpital parce que dans l'argument, il avait est un point essentiel, c'est la capacité pour ces jeunes médecins d'avoir un un lien privilégié avec l'hôpital de proximité et je crois que on n'a autant travaillé d'employer de santé sur ce lien hôpital avec l'implication du directeur de l'hôpital qui a fait quelque c'était des jeunes médecins qui avaient un choix un panel d'installation et l'autre sujet qui concerne tous les les élus locaux, c'est qu'on a passé beaucoup de temps à parler finalement non pas de médecine, point de santé mais a parlé d'attractivité du de du territoire de la commune et de l'environnement familial, on a passé beaucoup de temps à parler de de d'emploi notamment pour pour les conjoints, on a passé beaucoup de temps à parler de service public dans la commune, notamment comment elle que faire pour les enfants pour la scolarité pour la garderie et finalement dans les dialogues qu'on a pu avoir, je pense que c'est l'ensemble de ces arguments qui a fait basculer le choix, mais vraiment, je pense que les élus locaux, même ce n'est pas des spécialistes, on a un vrai rôle et puis un projet de maisons de santé ou de Pôle santé s'la fois naturellement avant tout le projet de santé mais c'est tout, certains environnements qui crée un moment donné, des conditions favorables dans des territoires qui apprenait à vue n'avait pas des grands atouts, ni au bord de la mer d'à côté des grandes, des grandes villes, mais je pense que c'est l'énergie collective qui a fait basculer et la création de cette maison de santé qui fonctionne très bien aujourd'hui. Merci, Madame Cohen vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le le président je pense qu'on est, on est tous d'accord et on est en en recherche de solutions pour essayer de régler le problème et tous les secteurs connaissent des déserts médicaux, ça je crois que c'est vraiment très important de le dire parce que souvent l'image, c'est quand même déserts médicaux, donc c'est en zone rurale, mais en zone urbaine Madame le ministre a dit Paris mais effectivement, Paris et toute l'Île-de-France connaît dans sa certain nombre de de de quartier ces problématiques là, donc ça concerne vraiment tout le monde, moi je suis très dubitatif, même si je comprends mes collègues qui sont recherche de, de, de, de solutions sur la proposition, la proposition faite, pourquoi, parce que je trouve un petit peu curieux de penser donc au déconventionnement des médecins qui, pour moi, va toucher le patient.

mais là, quand on dit que les médecins ne vont pas être conventionnés si, si, ça veut dire que donc le patient qui a le libre choix de choisir son médecin, à ce moment-là en subira les conséquences parce qu'il y aura pas de remboursement je ne vois pas pourquoi on fait reposer sa sur sur le patient, c'est pour ça que je suis, je suis dubitative plus les les raisons que Catherine Deroche a longuement

Bien, merci, je considère que les explications de vote ont eu lieu sur l'ensemble de ces amendements, il y a encore Madame pas Fillinger. J'ai il y a pas de problème assez ouvert la nuit, on ouvrira lundi on peut continuer sur cet amendement encore donc Madame Schillinger et et monsieur d'accord à vous. j'ai apprécié dès le le dit. De madame de roches et puis de madame la ministre, je vous, je voulais vous dire que moi je suis dans un territoire où il y a des médecins, mais seulement c'est l'organisation des lieux où sont les médecins, nous avons 3 médecins qui sont partis d'une ville de de 7000 habitants pour rejoindre ma commune qui a 3400 habitants, il n'avait pas besoin de partir, ils étaient à un kilomètre, donc moi je pense que disent les élus font des efforts dans tous les territoires pour trouver des établissements pour vraiment trouver les le lien qu'il faut même proche des hôpitaux mais je là où je je vois qu'il y a un manque c'est les relations qu'ont les médecins entre eux ils ne discutent pas entre eux, ils ne se projettent pas entrent dans un territoire où il y a souvent 30 médecins sur j'ai pas de 30 kilomètres à la ronde, il ne s'il n'est, il ne oui mais même s'ils sont libéraux, ils ont un devoir d'organisation Mali il y a des hôpitaux, il y a des spécialistes, il y a des moyens de garde et je pense que c'est là où il faut trouver un référent qui les met en lien, parce qu'il faut passer outre des égo et des des uns et des autres, mais je crois qu'aujourd'hui c'est vraiment cette politique qu'il faut mettre en en route pour que ces Liens se fasse,

j'ai apprécié moi que Madame la Ministre, présente un plan qui soit une sorte de bouquet toutes ces idées qui, on le voit marche ici marche moins bien dans le département voisin,

il y a un monsieur désert médical ou une personne, une dame bien sûr, une personne qui soit chargé de ce management, ça management de projets dans les entreprises quand vous avez une idée comme ça, nouvelle ou un problème majeur qui se pose, on ne peut pas le résoudre, individuellement, on voit bien que chaque maire aujourd'hui chaque président de syndicat chaque président de communauté essaye de trouver la solution, mais il n'a pas le référent qui possède les clefs en quelque sorte pour pouvoir le guider dans une bonne pratique et il se trouve isolé, donc ce que je suggère, Madame la Ministre, c'est que il y a un manager de projets dans chaque ARS chargés de porter et surtout d'animer le territoire pour apporter à chaque élu la solution ou les solutions qui lui paraissent la meilleure des meilleurs. Merci, Monsieur Vasseur Monsieur le Président Madame je crois, j'ai pas eu le temps de de trop calculé, mais c'est plus de 120 ou 130 sénateurs qui ont qui ont signé ces différents amendements donc ça correspond quand même à

et je voudrais dire aussi que je vais pas raconter ma vie, mon épouse est médecin, donc je suis aussi dans un milieu médical et lorsqu'on en parle sur nos territoires, beaucoup de médecins isolés ment ne sont pas du tout hostile au fait de

je crois qu'il y a néanmoins des zones surdotées en France même si personne n'a levé la main il y a quand même des endroits en France où on sait que, il y a un nombre de médecins conséquents, c'est un peu incompréhensible de continuer à ne pas vouloir faire en sorte de de d'abord privilégier les secteurs qui ne sont pas sur-dotée par rapport au secteur surdotées alors que c'est des médecins conventionnés que c'est des actes qui sont pris en charge en totalité, je, je, je, je voulais dire, donc moi je ne peux pas retirer les amendements, alors qu'on est, je crois, 80 ou 90 de notre sensibilité à l'avoir signé, puis 130 ou 140 au total.

madame la ministre, moi je voudrais intervenir sur le plan de de la logique en tant qu'enseignant et par rapport à ce qui se passe à l'université parce que finalement il y a des rapprochements à faire qui sont intéressants, nous manquons de façon criante d'enseignants dans tous les niveaux et votre gouvernement va instaurer, par le biais de la sélection, vous l'appelez pas comme ça, mais ça revient la même un numerus clausus qui n'existait pas à l'université, par ailleurs, dans les études médicales, ma fille en fait donc je, je, je vois ce que je vois ce que c'est, aujourd'hui, en première année, il y a un taux d'échec de 90

la pénurie, par des politiques malthusiennes et je ne comprends pas comment on peut gérer des pénuries, à la fois d'enseignants et de médecins en restreignant l'accès aux études, à la fois de médecine et aux études générales merci.

actuellement il y a beaucoup de médecins ce qu'il a dit, René-Paul Savary, mais il y en a 25 pourcent qui ne s'installe pas ou qui ne remplace pas, donc moi quand j'ai signé Ceuta moment je ne pensais pas qu'il est vraiment une contrainte énorme puisque c'est la RS qui défini les zones surdotées et c'est uniquement dans ces zones à titre expérimental que on peut voir si cette petite coercition effectivement peut apporter quelque chose, alors bien sûr, je pense que, comme ça a été dit que l'article 35 va nous apporter des solutions merci. Merci, alors Monsieur le président Millon et Madame la Ministre, ensuite à demandé à nouveau prise de parole. Oui, merci Monsieur le Président, je vais pas moi revenir sur tout ce qui a été dit, parce que je suis d'accord avec tout pays tout le monde finalement un petit peu raison mais attends, t'entends je je vais, je vais revenir sur 2 ou 3 choses : il me semble que l'important quand même, et ça a été dit, avant hier, ça a été dit, aujourd'hui aussi, c'est évidemment l'attractivité des territoires et l'aménagement du territoire qui permettent dès à dès, médecin de venir s'installer, alors je voudrais surtout adressé à ceux qui ont signé ce amendement en prenant l'exemple inverse en vous demandant d'imaginer le ressenti des médecins qui sortent de la faculté de médecine et qui voient ce genre d'amendements apparaître votées par notre assemblée ou voté par l'Assemblée nationale, mettez-vous à la place de ces gens-là et imaginez leur ressenti, et pour que vous puissiez imaginer le ressenti, je vais vous faire l'inverse, je suis dans une zone sous-dotée en entreprise, donc je présente un amendement qui interdirait aux chefs d'entreprises de s'installer dans les zones surdotées en Île-de-France ou dans Les Hauts de Seine, par exemple, et je dirais simplement bon, va pour que ces entreprises ne s'installe pas là où il y a déjà beaucoup d'entreprises ont remédié SF en classe pour les entre chefs d'entreprise concernées on remet les cotisations sociales en place pour les entreprises ainsi concernés qui s'installeraient dans des zones surdotées et on double les impôts parce qu'elles s'installent dans les zones surdotées, c'est exactement la même chose que vous ce que vous voulez faire avec le médecin, ce serait ça pour les entreprises qui s'installera aux zones surdotées, regardez bien votre ressenti et dites-vous bien que ce ressenti se fait aussi pour les médecins, pour les étudiants en médecine et que dans ces conditions, ça les empêchera peut-être d'aller dans le vers la médecine d'aller ailleurs. Merci Monsieur le Président, Madame la ministre. Je souhaitais répondre sur le numerus clausus, puisque vous m'avez interpellé et vous avez raison, je pense que c'est dramatique, une classe d'âge qui sont, en général, en plus des étudiants assez brillant avec des mentions très bien au bac soit refoulés comme ça des études de médecine avec un numéro clausus très sévère, la raison de ce numéro que jusqu'on a connaît je, je l'ai dit je crois 1er jour c'est que on n'a pas trouvé d'autre moyen pour réguler l'augmentation des dépenses de santé que le numerus clausus. Parce que les médecins sont payés, ça été un raisonnement. assumer de différents gouvernements depuis 30, 40 ans, avec une mauvaise anticipation effectivement de la conception de la vie professionnelle qu'ont les jeunes aujourd'hui, je ne parle même pas de la féminisation, mais qui fait qu'aujourd'hui non seulement quantitativement, nous n'avons plus assez de médecins, et qualitativement, ils n'ont pas envie de la même ville vie que celle des médecins d'antan, dont acte, maintenant ce constat ont été fait par quelques gouvernements antérieurs le numerus clausus a été un peu augmenté, il est passé de 6000 à 8000 étudiants non plus 25

de leurs études et de leur internat puisqu'ils sont tous à l'internat maintenant dans 12 ans donc en 2030. Nous aurons et nous le savons, une démographie médicale qui aura d'ores et déjà augmenter par rapport à ce qu'elle est maintenant nous savons que nous à vaincre en 2025 et que, en 2030, nous aurons une démographie médicale supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui, donc si nous ouvrons numerus clausus largement en 2018 jusqu'en 2025 vont sortir un nombre de médecins très important entre 2030 et 2035 et donc nous aurons exactement inversé ce que nous subissons aujourd'hui, c'est-à-dire une démographie médicale négative, donc nous avons intérêt collectivement à nous interroger sur quel sera l'exercice de la médecine en 2035 de combien de médecins nous aurons besoin, quel sera l'exercice coordonné entre professionnels, quels seront les démographie des nouveaux professionnels avant tout simplement d'ouvrir les vannes du numerus clausus parce que nous, nous allons à une catastrophe dans l'autre sens, avec énormément de médecins et si nous poursuivons en plus une tarification à l'acte, ça ne sera pas un Ondam à 2,3 pourcent qu'il nous faudra un, ce sera un Ondam à 7 pourcent soyons clairs, hein, parce que la régulation de la tarification de la médecine de ville, aujourd'hui elle est compliquée, donc d'une part je souhaite modifier un peu la tarification tarifications des médecins en n'associant à la tarification à l'acte, une tarification à la qualité à la pertinence, ça permettrait par exemple de réguler ce que vous appelez les sur zones surdotées où on considère que des médecins en grand nombre étant étendant ils font beaucoup d'actes dont certains sont inutiles, c'est la raison pour laquelle je souhaite travailler sur la pertinence des actes et la régulation par la qualité et la pertinence, ça permettra donc dans des zones soi-disant surdotées à ce qu'il y a un peu moins d'actes répétitifs et pour moi c'est une bonne régulation par la qualité plutôt que par la coercition je souhaiterais rajouter de la tarification à la qualité à la pertinence, ce qui nous permettrait éventuellement d'augmenter le nombre de médecins mais à ce moment-là de façon réfléchie et en ayant une projection de ce que va être la médecine en 2035, donc c'est une réflexion que nous allons avoir dans les années qui viennent avec les PLFSS successifs, mais je pense que, à la fois la régulation Commercy tive à la fois l'augmentation du numerus clausus, ce sont des idées, à mon avis un peu simple par rapport à la complexité du problème et donc c'est la raison pour laquelle je je ne suis pas du tout favorable à ces amendements. Merci pour cette toute petite intervention. Je je j'ai notre assemblée, nous avons fait peut-être tout à l'heure sera fera 8 mai 3 amendements une vous projetez une ouverture lundi. à ce rythme, c'est pour ceux qui veulent anticiper, donc nous allons passer au vote 4, 2, 3 amendements identiques puisque un n'a pas été défendue 207 rectifier quater 421 rectifier bis, et le 560 rectifier. Qui pour.

Qui est pour. Qui s'abstient, il n'est pas adoptée ensuite les 391 rectifier bis. Qui est pour.

493 rectifier Madame Cohen, vous avez la parole. Merci Monsieur le le président donc dans la la prolongation et de l'amendement qui a présenté Dominique Vatrin et on fait du débat que que nous devons avoir, nous faisons donc un autre. Amendement qui est de de fixer des critères pour ce zonage et de soumettre l'installation des médecins à l'autorisation des ARS dans des secteurs sur Dudus densifier pour certaines spécialités médicales. Afin justement de pouvoir, je m'en emmêle dans les papiers afin d'éviter que certaines zones soient mieux pourvus alors que d'autres manquent cruellement de médecins, je rappelle, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises que il y a, il sait aussi qu'une question d'actes attractivité territoriale et de maintien ou pas d'un haut niveau de service public, sur le territoire, je crois, et nous l'avons tous plus ou moins dit que le critère financier secondaire dans le choix d'installation d'un professionnel de santé qui regarde en priorité à exercer près d'un établissement hospitalier, ça je le redis, fortement notamment ainsi à dans un cadre où il va pouvoir travailler avec d'autres collègues dans une pratique plus partagé, que ce soit d'ailleurs dans un centre de sang. Ou dans une maison de santé et puis bien sûr, il recherche aussi à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, d'où l'importance aussi de développer des services publics, on a dit que la la situation était grave, moi je voudrais quand même parce que je crois que Madame la rapporteur l'a rappelé, mais finalement c'est bien d'parfois la répétition, c'est très pédagogique, la mission de la MNEF, hein, qui a été conduite donc par Jean-Noël Cardoux et Yves Daudigny promouvoir l'innovation santé dans les territoires et qui dit que la densité médicale devrait connaître un plus bas historique à 3 médecins par habitant en 2023. Donc il faut effectivement, compléter les mesures qui ont été énoncés par Madame la ministre, nous pensons que notre amendement est de nature à aider. Madame Cohen, l'avis de la commission Madame la rapport. Alors les zonages qui Servent de base à l'attribution des aides à l'installation des professionnels de santé dans les zones sous- dotées font alors actuelle l'objet de d'une révision qui est construite en région par les ARS, vous avez dû le vivre dans vos dans votre département respectif afin de mieux objectiver les besoins de l'indicateur synthétique a été développé et la commission n'a pas trouvé opportun de fixer dans la loi de nouveaux critères, c'est donc une demande de retrait ou un invité favoris. Merci la vie du gouvernement défavorable. y a-t-il des explications de vote, il y a une demande de retrait non vous maintenez donc on passe au vote qui est pour. Est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adoptée, donc nous passons maintenant, après l'article 35 à l'amendement 157 rectifier. Monsieur. William si président le décret 2000 16397 du 12 octobre 2016 relatifs aux conditions de délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices et aux règles d'exercice de la profession d'opticien lunetier donne la même durée de validité de l'ordonnance médicale pour la primo-délivrance de l'équipement optique ou son renouvellement, il peut par conséquent se poser le cas de la délivrance de produits optiques avec une ordonnance anciennes de plusieurs années, laquelle n'aurait pas été utilisé initialement or lors de la première délivrance l'opticien lunetier ne pourra pas adapter la prescription initiale, c'est bien lui et seulement permis lors du renouvellement de l'équipe de optique si l'ordonnance est encore valable

il est proposé que la possibilité de prise en charge par l'assurance maladie pour la première délivrance soit limitée à la première année suivant l'établissement de l'ordonnance afin de limiter le risque de dépenses inadapté pour l'assurance maladie, ces mesures n'amèneront pas de charges supplémentaires pour l'assurance maladie et sont sans conséquence sur les possibilités de renouvellement et d'atomisation des ordonnances par les auditionner elles amènent une clarification nécessaire pour une meilleure pertinence dans le parcours de dérive de délivrance et de renouvellement des équipements optiques merci. Merci madame la rapporteure votre avis. Alors on aborde la 2 amendements, enfin on verra ça tout à l'heure où les 12 sur la filière visuelle, on a. J'ai évoqué le sujet hier puisque certains amendements étaient présentés après l'article 35 la filière visuel, elle s'est elle s'est organisée il y a eu dans les les mois qui ont qui nous précèdent, vraiment un équilibre qui a pu être trouvé, même s'il n'est pas encore totalement abouti dans certains sur entre les ophtalmologistes les orthoptistes et les opticiens, chacun ayant des missions bien bien défini et et avec des degrés de de compétences sur certains sujets différents. Mais il y a quand même eu un travail qui a été fait de façon à pouvoir faire en sorte qu'il y ait un accès que les ophtalmologistes dont on sait la difficulté parfois et la la durée pour avoir un rendez-vous puisse avoir des tâches qui soient effectués par les orthoptistes sous leur responsabilité ou ou aussi un travail

pour l'accès aux équipements ça c'est c'est relativement, relativement simple sur le fond, moi je suis pas opposé à l'amendement que vous proposez parce qu'en effet il y a une sécurité dans les être devait être noté, il faut même si une prescription de lunettes paraît simple, ce qui est important aussi c'est le le dépistage de de pathologies oculaires qui pourrait évoluer à bas bruit et il faut qu'il est, puisse y avoir dans ces cas-là, retour à Tanger, mais vu le travail fait par les,

qu'ils vont pouvoir se se décliner au début de l'année 2018, donc c'est une demande de retrait. Simplement sur un seul amendement. Oui, pardon, je, je pense que cet amendement durcit les conditions d'accès en fait aux équipements d'optique et donc ça ne va pas dans le sens d'un accès plus facile aux soins je suis défavorable.

Monsieur Amiel, vous avez la parole. avait porté sur la capacité de renouvelle ses équipements de lunettes sans passer par une consultation chez un ophtalmo, si rien ne remplacera l'action du médecin dans la prévention, le dépistage et le traitement des maladies visuelles, les difficultés actuelles pour obtenir des rendez-vous chez ces professionnels ne sont pas sans conséquences pour les citoyens, il est ainsi proposé que, sauf contre indication médicale signaler les orthoptistes qui pourront dès le 1er janvier 2018 procéder à l'acte de mesure de l'acuité visuelle et de la réfraction puissent, au même titre que les opticiens renouveler en fonction de ces résultats, les prescriptions de lunettes et ou de lentilles. Oui, madame la rapporteure votre avis. avis. Sur cet amendement, c'est une demande de retrait ou un avis défavorable, ça rejoint ce que j'ai dit précédemment et puis l'orthoptiste, c'est quand même un métier métier différentes, souligne l'opticien, donc je ne suis pas favorable. Mais, madame la ministre avait du gouvernement. Oui monsieur la mienne votre amendement propose aller plus loin, de donner aux orthoptistes les mêmes prérogatives les opticiens, cela pourrait être envisagé, mais nous sommes vraiment nécessaire de concerter les professionnels avant donc je vous propose un retrait.

Merci monsieur le président, un amendement qui me tient particulièrement à coeur, Madame la ministre un pourrait et essayer de gagner du temps dans le le traitement des troubles neuro-dégénérative, tout à fait essentiel, y a une impatience des patients à un nombre important bien entendu et puis une impatience aussi des biotechnologies qui n'ont pas forcément les moyens parce que c'est un investissement de trop long terme qui fait que les investisseurs, là aussi, ne se précipitent pas forcément contrairement à des biotechs investissent dans dans d'autres domaines, donc il s'agit de gagner du temps administratives à travers une autorisation différentes qui n'existe pas aujourd'hui mais qui rentre dans le droit européen qui serait l'utilisation testimonial éclairée et surveillée alors pourquoi testimonial parce que c'est une implication : une responsabilité du malade qui désirent par instinct de survie, prendre le le risque de d'améliorer sa maladie à travers des médicaments qui n'ont pas au jour d'aujourd'hui, par définition encore suffisamment montré leur efficacité, il y a un véritable risque c'est la différence par rapport au compassionnel bien sûr parce que c'est véritablement un choix du malade qui prend cette responsabilité, donc il faut que ils soient bien entendu complètement conscient des des risques encourus et surveiller, parce que il y a effectivement la vie Vicky étant en jeu et nous avons ces organismes tels que l'ANSM qui fait fort bien son travail, que je tiens à remercier, elle a participé, entre autres, à la rédaction de 7 ans cet amendement de façon très volontaire et se trouve que c'est très important, donc faut une surveillance il mérite peut-être d'être encore améliorée, ce sera peut-être le but de la discussion avec l'Assemblée nationale, mais je pense que son but ultime, c'est véritablement gagner du temps, on gagne quelques années dans ce domaine-là, grâce à cette avancée administrative, je crois qu'on sera tous honorés d'avoir participé à cette décision. la Commission a été sensible à l'objectif qui est d'accélérer la mise sur le marché une molécule innovante dans dans le domaine qui est celui des troubles neuro-dégénératif dans lesquels les les évolutions sont lentes à en il y a beaucoup d'innovations en matière de donc mais c'est vrai que dans ces domaines qui, qui sont des pathologies douloureuses, avec des conséquences sociales et et et sanitaire lourde, là il y a une opportunité peut-être de d'accélérer l'accès à l'innovation et la la Commission émis un avis favorable. L'avis du gouvernement, Madame la Ministre. par rapport à l'instruction, donc on a pu faire de ce dossier parce que je vois quand même quelques petits risques, notamment le risque de mettre à disposition de patients des médicaments qui auront été très très peu évaluer avec des risques évidemment d'effets secondaires, donc c'est la raison pour laquelle, en général, on préfère des essais cliniques à des mises sur le marché très précoce ou des remboursements très précoce, d'autre part, vous proposez, que ce soit pas pris en charge par la sécurité sociale, donc qui hyper ce que ce serait les patients les patients, ça fait une médecine à 2 à 2 vitesses, donc je pense qu'il faut qu'on y travaille encore, je pense qu'il y a un sujet effectivement pour des maladies rares et donc je vous propose un retrait et ne retravailleront ce sujet éventuellement avec vous si vous souhaitez. Monsieur Savary. Oui, madame la ministre, je comprends tout à fait, bien que vous avez besoin de sens mais je crois que, de temps, pardon, mais qui sont aujourd'hui sur les paillasses des laboratoires et le temps pour lequel qui sera nécessaire pour qu'elle se retrouvent sur les étagères des pharmacies, il y a beaucoup de patients qui seront, d'ici là dans leur situation, avec un coût sociétal particulièrement important si les autorisations actuelles permettaient de gagner du temps, effectivement, on pourrait les, les, les, les, les, les prendre et et s'en servir, il y a une différence, Madame la Ministre, effectivement, entre le compassionnel et le testimonial ou dans le compassionnel effectivement et c'est prévu dans l'ensemble des atténue reconnue sur le plan européen, il y a effectivement une prise en charge normale à ce moment-là, qui est pris en compte et c'est un extrait c'est gratuit le testimonial effectivement est un acte volontaire de prise de risque du malade et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas l'empêcher de payer, il risque sa vie et peu risqué aussi de financer les propres médicaments nécessaires à l'amélioration de sa santé et Servent de témoignage pour d'autres malades et en sauvé à l'avenir, c'est véritablement une innovation du XXIe siècle, c'est pour ça que j'ai souhaité que ce soit l'article 35 il mérite sûrement d'être approfondie mais je ne retirerai pas parce que je pense que si on arriverait si on par le biais des décrets derrière nous arriverions bien sûr à garantir la gratuité de l'accès des soins, c'est tout à fait important mais il faut également que celui qui souhaite investir puisse intervenir, c'est là qu'il faut trouver l'articulation nécessaire, il va plus que des soins, c'est de la survie, donc on doit trouver une égalité de tous pour accéder à cette rue survit dans ce domaine des troubles neuro-dégénérative, c'est la raison pour laquelle je demande à mes collègues de voter unanimement encore cet amendement comme ils l'ont fait à la commission des affaires sociales de façon à avancer dans la réflexion. Bien, donc nous allons consulter notre assemblée, il y a un avis favorable de la commission, un avis de retrait et donc défavorable du gouvernement. Est pour.

les actes de téléconsultation de télé-expertise en les sortant du cadre expérimental dans lequel ils étaient. Monsieur, vous êtes en train de parler de d'autres choses de ce 28 rectifier, allez on on va dire qu'il est défendu de 228 quater l'avis de la commission. la commission avait été favorable lors de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2017 à la mise en place de l'Avantage maternité pour les médecins, elle avait même souhaité l'étendre à tous les médecins sans le restreindre selon leur mode au lieu d'exercice une avancée similaire pour les autres professionnels de santé sur un progrès social, en particulier dans des métiers fortement féminisée, c'est donc un avis favorable. Donc, avis favorable, l'avis du gouvernement, Madame la ministre. Défavorable. Nous allons voter, qui est pour. Ce qui est contre. Qui s'abstient-il être adopté, nous passons à l'article 35 bis. Amendement 119 de madame la rapporteur Madame Europe, vous avez la parole. Oui, cet article a été inséré à l'Assemblée nationale et prévoit la remise d'un rapport au Parlement Latif aux dépenses des indemnités journalières au type de la maladie de leur articulation avec les dispositifs de prévoyance, c'est vrai que le sujet important contenu la dynamique de cette dépenses qui représente, pour le seul régime général plus de 7 milliards d'euros en 2016 en progression de 5 pourcent sur un an, des économies sur ce poste Somerset j'attendu pour 2018, un objectif de maîtrise des dépenses, relevé de 100 à 160 millions d'euros par le président présent Plfss il appartient notamment la CNAM de tenir cet objectif, est d'engager des actions de faire des propositions, il nous a semblé qu'un rapport supplémentaire sur ce sujet ne fera pas avancer les choses, d'où cet amendement de suppression de l'article. L'avis du gouvernement, Madame la Ministre. Sa jeunesse, je ne vois pas de demandes de parole, donc nous allons voter, qui est pour. Qui et contre qui s'abstient. Cet amendement était adopté, ce qui supprime l'article 35 bis, l'article 36, maintenant il y a des paroles sur l'article d'abord une parole monsieur

une plainte pour distorsion de concurrence, après la diffusion d'une campagne publicitaire réalisé par une mutuelle pour des téléconsultations, Madame la Ministre, la publicité, précise que ce service est gratuit pour ses adhérents et dans le cas contraire, ce sera évidemment payant cet exemple montre l'importance que prennent les mutuelles, organismes complémentaires ou assurances en matière de soins alors que ce n'est pas leur rôle, la médecine n'est pas un commerce, nous savons tous les sous couvert de donner un meilleur accès aux soins ces organismes sélectionnent leurs patients qui seront évidemment captifs, pouvez-vous, Madame la ministre, nous donner l'avis du gouvernement sur ce type d'action. madame la ministre, vous voulez aussi répondre à Monsieur le Président, ou attendent des amendements

Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, donc la pharmacie d'officine établies dans ces territoires isolés doit pouvoir mettre au qu'en contact au sein de son espèce de confidentialité, le patient avec son médecin traitant ou le service hospitalier lorsque cela est nécessaire, la pharmacie de officine est une espèce de santé réglementé qui peut utiliser des outils de télésanté pour renforcer les Liens entre les médecins et les populations éloignées aussi, il est essentiel que la convention pharmaceutique prévue à l'article L 162 tiré cesse tiré du code de la sécurité sociale soit intégrée dans cet article, permettant ainsi la prise en compte du rôle des pharmaciens dans le développement dans certains territoires de la télémédecine. Merci. La commission a trouvé légitime en effet de reconnaître le rôle des pharmaciens dans le déploiement de la télémédecine, elle a émis un avis de sagesse. Merci madame la Ministre votre avis. Une réflexion sur l'évolution des compétences des pharmaciens d'officine et est d'ores et déjà engagé avec l'assurance maladie dans le cadre conventionnel et nous avons, de toute façon dans les actes de télémédecine déjà acté que les pharmaciens peuvent participer aux actes de télémédecine, puisque c'est aussi vrai pour d'autres professionnels de santé, comme les infirmières qui vont participer aussi aux actes de télémédecine quelque part cet article comprend les pharmaciens. Donc la rédaction proposées dans l'amendement ne nous paraît pas juridiquement satisfaisante, nous vous proposerons un amendement gouvernemental de 597 qui permettent de d'avoir une rédaction plus satisfaisante donc je vous propose un retrait en faveur du de l'amendement 597. Je me tourne vers Madame Moret Richaud, vous vous propose un retrait vous le maintenez sur le maintien. Il est maintenu, donc il y a une sagesse de la Commission, il y a un non du gouvernement qui est pour la attendez attendez madame le rapport. Oui, je comprends que que notre collègue intéresse amendements mais c'est vrai que l'amendement du gouvernement qu'on avait pas vu n'avait vu n'avait pas examiné en commission répond de façon aux mêmes objectifs, mais de façon juridiquement mieux mieux formuler mais c'est vrai qu'on avait passé en commission, je comprends que vous me bien je pense que ce serait préférable, à ce moment-là de le retirer. Bien, donc je me retourne à nouveau après ce conseil de Madame la la rapporteure vers vous. Au vu des explications de Madame le le rapporteur, effectivement je retire l'amendement. C'était les les mêmes que celles que les explications de Madame la Ministre, mais nous allons donc passer à l'amendement numéro 120.

Nous passons au 386 rectifier bis. Monsieur, vous avez la parole. Merci monsieur le président, ministre d'amendement a pour but de mettre un peu de souplesse en remplaçant le mot vidéo transmission par les mots technologies l'information et de la communication, en effet, l'exigence de la vidéo transmission pourrait aboutir dans certains cas et dans certains territoires un échec technique du fait de l'insuffisance de de réseaux adaptés chez le patient ou lors de ses déplacements cette conditions créer une rupture des qualités, notamment pour les personnes âgées ou les ménages les plus modestes qui ne sont pas, qui ne seraient pas équipés de type de le vidéo-transmission et qui ne pourraient pas accéder à ce nouveau bien, c'est pour ça que le présent amendement atténue le caractère impératif et systématique de tu politisation de la vidéo transmission pour les actes de téléconsultation et la rédaction ici proposé demande de la souplesse permet ainsi de garantir les actes de téléconsultation une population plus large: quel que soit son territoire merci. Si monsieur opère l'avis de la commission Madame. La porte, je comprends ce que. Que propose Monsieur opère néanmoins la vie de retransmission garantit une certaine qualité de soins, et au vu de la rédaction de proposer, on pourrait penser que c'est un simple appel téléphonique, donc la commission a préféré s'en tenir à la rédaction proposée. Madame la Ministre défavorable, défavorable, il y a-t-il des explications de vote, je n'en vois pas donc. Avis défavorable de la commission avis défavorable du gouvernement qui est pour cet amendement.

Monsieur derrière au à la parole. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, l'article 36 prévoit de développer la télémédecine, afin d'éviter les fraudes, notamment, il convient d'encadrer la manière dont les prescriptions issus des téléconsultations seront transmises aux pharmaciens de façon à ce que cela soit sécurisé, en effet, à la faveur de ces nouveaux développements, les patients présenteront leurs ordonnances par des moyens électroniques divers exemples les smartphones en décalage avec les textes existants, qui prévoit que le patient doit présenter l'original de l'ordonnance l'introduction de la notion d'ordonnance dématérialisée dans le code de la santé publique permettra par ailleurs de poursuivent la logique jusqu'au bout en dématérialise en tout le processus de la consultation à la prescription, voilà le l'objet de cet amendement. madame la rapporteur. Vrai que l'enjeu de la dématérialisation des prescriptions dépasse le Champ de la thématique, même si les pratiques, comme l'a dit notre collègue vont se développer avec les téléconsultations alors la précision demandée peut paraître redondante avec les dispositions qui siège à prévues en matière de transmission des données de santé toutefois l'amendement, a le mérite de poser les enjeux, notamment pour prévenir les risques de fraude et la commission a émis un avis de sagesse.

Explications de vote Monsieur Deriot. Oui, bien écoutez mon jeu d'entendre Madame la rapporteur et madame la ministre, si les conditions de sécurité sont déjà à vous assurer, je retire effectivement l'amendement.

Toujours bien sûr, merci Monsieur le Président, la Ministre cet amendement propose de d'un associé, les professionnels de santé, médecins mais aussi pharmaciens aux ou infirmiers aux travaux permettant le déploiement de la télémédecine via leurs représentants syndicaux et Ordinn l'intégration dans le droit commun tarifaire de la téléconsultation est une excellente option pour autant il est indispensable que cette thématique nouvelle créatrice de lien renouvelé entre la ville et l'hôpital au service des parcours de soins et de vie des patients à domicile associe d'emblée tous les professionnels de s'emporter, qui pourront être concernés par les nouvelles dispositions de l'article L 162 14 Merci le 242 rectifier coacteur Madame Delmont-Koropoulis. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mais, chers collègues, l'article 36 de ce PLFSS vise à intégrer dans le droit commun tarifaire certains actes de télémédecine, c'est-à-dire la télé-expertise et la téléconsultation, réalisée par vidéo-transmission il maintient un cadre expérimental pour les seuls acteurs de télésurveillance, la télémédecine constitue un des leviers que nous devons activé pour lutter contre la désertification médicale dont souffrent, tourner des 2 territoires si la télémédecine est loin d'être la seule solution à proposer pour renforcer l'accès aux soins, sa démocratisation, aura un impact significatif pour nombre de nos concitoyens, notamment pour ceux souffrant de pathologies rares et traitées par un nombre restreint de praticiens en cela la fixation d'une tarification de droit commun, des actes de télémédecine par les partenaires conventionnels constitue une bonne option, car comme l'ont souligné les rapporteurs dans heure est aux examens, des articles, la commission a depuis longtemps identifié la tarification de droit commun, des actes de télémédecine comme une condition préalable préalable à son réel déploiement, la création d'une commission de télémédecine auprès de l'Union nationale des Caisses d'assurance-maladie prend donc tout son sens, il est indispensable que cette thématique nouvelle créatrice de lien entre la ville et l'hôpital au service des parcours de soins et de vie des patients à domicile à ceci: les représentants des médecins libéraux, les professionnels hospitaliers : les fédérations hospitalières représentative des établissements publics et privés, les représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance-maladie et les représentants de l'Union nationale des organismes, des caisses d'assurance maladie complémentaire, ce dispositif est pas par ailleurs établi en analogie avec l'article L 162 du code de la Sécurité sociale, introduire l'article 99 de la loi de frs FSS pour 2017 et qui a créé une commission des équipements matériels lourds d'imagerie médicale, je vous remercie. Et Madame amendements identiques Monsieur Daudigny. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, l'amendement identique, je ne comprends pas les arguments déjà explosé fort bien par mais collègues je rappelle par contre mon soutien, qui avait déjà lui aussi était exprimé vos articles 35 et à l'article 36 la proposition vient donc en appui de cette intégration dans le droit commun des actes de télémédecine téléconsultation excellente option est certainement une ouverture considérable pour ses activités avec toutes les observations qu'elles vont certainement amené dont celle qui a été donné à l'assistance, il y a quelques instants par monsieur le président de la commission des affaires sociales, le débat en même temps est ouvert entre le rôle des Nations de l'assurance-maladie et des organismes complémentaires, il faudra remonter dans notre histoire récente pour comprendre pourquoi aujourd'hui nous avons cette dualité aussi forte qui a été un moment marqué par la création de l'Unocal, c'est-à-dire de l'Union des organismes complémentaires d'assurance maladie, je vous remercie.

Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie, nous l'avait largement évoqué lors de l'audition, alors il semble qu'il n'y aura pas lieu prévoir à ce stade des modalités dérogatoires par rapport à la fixation des autres tarifs conventionnels alors les auteurs des amendements s'inspire du modèle de la commission des équipements matériels lourds qui en fait en effet des enjeux particuliers pour les établissements qui exploitaient ces appareils ces apparaît alors sur ai le sujet de la thématique mais il sera néanmoins important, en effet, d'associer l'ensemble des acteurs en ville et à l'hôpital et c'est l'idée qui sous-tend ces amendements, la commission a donc souhaité connaître l'avis du gouvernement. Madame la ministre, votre avis alors. Résidant c'est l'article 36 c'était une demande de tout le monde que la télémédecine rentre dans le droit commun et puis se déployer rapidement, donc il y a une forme de contradiction à vouloir créer une commission qui ralentirait les procédures d'inscription dans le droit commun, on a considéré dans cet article 36 que les actes de télémédecine, devait être discuté dans le cadre. Conventionnel comme toute acte médical, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une réflexion avec les établissements de santé, pour voir comment ils s'intègrent dans le dispositif, on a d'autres méthodes pour cela, on a la tarification forfaitaire, la tarification parcours dans lequel on va pouvoir intégrer progressivement d'autres acteurs que simplement aujourd'hui la médecine libérale, qui fait l'objet de la négociation conventionnelle pour ces raisons, je vous propose un retrait sinon nous y défavorable, parce que nous ne souhaitons absolument pas ralentir le processus actuel mais bien entendu, nous allons discuter avec les établissements et tous les autres acteurs pour voir comment, progressivement on peut intégrer l'ensemble des acteurs dans les dispositifs de télémédecine de télé-expertise. Merci, il y a-t-il de l'explication de vote sur le 13 rectifier. Non, donc nous passons au vote. Alors il y a un avis défavorable, et le gouvernement a demandé un retrait, donc je ne fais je comprends effectivement l'explication qui a été donnée par Madame la ministre à dire dans un 1er temps je sois à l'intérieur de la convention, qui en fait la convention qui correspond à la convention médicale, donc avec les médecins, ça se comprend tout à fait, disons que ça a été un amendement d'appel pour ne pas oublier après l'ensemble des autres professions médicales comme en particulier, les pharmaciens, mais c'est vrai pour les infirmières qui elle voilà ah bah, écoutez, il faut bien vous êtes vous êtes combien de médecins par rapport à combien de pharmaciens, nous sommes ici, alors il faut bien que je sois celui qui, avec mes collègues, bien sûr que nous soyons ceux qui défendons la profession qui, je dois dire Rendez-vous bien compte et réfléchissez bien, si vous n'aviez pas le réseau des pharmaciens sur l'ensemble du territoire, il y aurait certainement d'autres problèmes, ça c'est à la suite de 25 ans de d'activité pharmaceutique et comme pharmaciens d'officine et comme pharmacien biologiste voilà donc je comprends effectivement ce que je vous demande, Madame la Ministre, mais vous l'avez précisé, c'est que dans un 2ème temps bien sûr, le pharmacien et autres professions soient associés, merci. Je, je, vous n'avez pas répondu à la question. Donc, l'amendement est retiré, nous passons maintenant aux explications de vote si on

Oui, cet amendement à la rédaction suivante, donc, l'article 36 de la présente loi de financement de la Sécurité sociale a pour objet d'habiliter les partenaires conventionnels à négocier avec l'Union nationale des caisses d'assurance-maladie, les modalités de réalisation et de tarification des actes de téléconsultation et de télé-expertise telle que définie à l'article L 163 61 du code de la santé publique, l'activité de télémédecine implique nécessairement une profession médicale, c'est pourquoi des négociations seront très prochainement ouverte entre l'assurance maladie et les syndicats de médecins pour intégrer la télémédecine dans la convention médicale dans un second temps, d'autres professions médicales ou non seront a amené à participer au développement de la télémédecine, notamment pour organiser l'accès des patients aux soins médicaux à distance, c'est pour cette raison que le projet de loi a d'emblée prévu une habilitation large impliquant l'ensemble des professions conventionnés, la convention des pharmaciens n'étaient pas incluses dans cet ensemble, il faut donc rectifier ce point et inclure les pharmaciens. Merci à l'avis de la commission madame la rapporteure. Je l'ai dit tout à l'heure, la, la commission n'avait pas pu examiner à l'amendement du gouvernement, mais lorsque j'ai demandé à Madame Moret réchaud de retirer son amendement profiter profiter du gouvernement c'était parce qu'il répondait en effet à cet oubli par rapport aux femmes. Eh bien, il n'y a pas d'explication de vote. Qui est pour. Qui est contre qui s'abstient-il être adopté, nous passons à l'amendement de 5 amendements en discussion commune. 231 monsieur Maurice et vous avez la parole. Oui, monsieur le président, madame la Ministre, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 mais fin au caractère expérimental de la télémédecine la généraliste pour partie en confiant aux partenaires conventionnels le soin déterminer les conditions de réalisation et tarification des actes de téléconsultation était l'expertise si l'objectif est de prévenir les hospitalisations et les transports de faciliter la coordination entre professionnels de santé et d'améliorer l'accès aux soins, il ne faut pas encore une expérimentation de 4 ans pour en faire de même pour la télésurveillance, celle-ci doit également entrer maintenant dans le droit commun afin d'être rapidement un outil au service des médecins et de leurs patients, je vous remercie. et les expérimentations qui pourront être menées pendant 4 ans grâce à l'article 36 donc du présent PLFSS ne doivent pas s'arrêter à la télésurveillance, la télémédecine doit également pouvoir permettre d'assurer le suivi du patient, telle est l'objet de cet amendement. Merci. L'amendement 121 rectifier de la commission Madame de roche. On on vise à préciser le Champ des expérimentations, des surveillances qui doivent concerner aussi bien les patients pris en charge en ville qu'en établissement de santé ou en établissement médico-social et procède donc à une coordination rédactionnel. 354 rectifier taire Monsieur Daudigny. Merci Monsieur le Président, Madame la ministre mais, chers collègues, je reste dans le domaine de l'insuffisance rénale chronique mais dans un autre cadre celui de l'article 36 la prolongation des expérimentations sur la télésurveillance est prévue dans cet article pour donc 2018 c'est expérimentation porte notamment sur la télésurveillance pour la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique mais n'intègre pas la dialyse péritonéale à domicile alors que bon, déjà derrière elle est pourtant nécessaire, on fait modalités de prise en charge du patient en favorisant son autonomie AT Gration, donc de la dialyse à domicile dans ces expérimentations paraît nécessaire pour éviter les ruptures de parcours de soins permettent de garder un lien avec le médecin hospitalier qui assure le suivi du patient et l'évolution de son mode de traitement, le cas échéant de cet amendement, je vous remercie. Merci, amendement 122 de la commission Madame le rocher. Grande de précision répond oui. Donc, votre avis sur l'ensemble des amendements qui vient d'être présenté. Alors sur le 231 cet amendement supprime l'expérimentation télésurveillance alors c'est vrai qu'on pourrait tenter de sortir, y compris pour la télésurveillance du cadre expérimental afin d'avancer vers une tarification de droit commun toutefois ce Champ paraît moins matures et pose notamment des questions assez complexe de prise en charge des dispositifs médicaux innovants sur lesquels, pour certains, on manque encore de recul, même si, paradoxalement, les expérimentations autorisées par la loi de financement de la Sécurité sociale en 2014 médecine sont les plus avancés en matière de télésurveillance plusieurs cahiers des charges ont été récemment publiés pour et passé un temps d'une insuffisance cardiaque, rénale ou respiratoire chronique, diabète ou porteurs de prothèses cardiaques, cela devrait permettre d'avancer, nous ne souhaitons plus rapidement dans les mois qui viennent, donc, sous réserve des assurances que ne donnera, Madame la Ministre, par rapport à l'avancement des expérimentations, des surveillants, ce serait une demande de retrait, mais nous demandons l'avis du gouvernement. Sur le 366 rectifier Bliss, d'après le décret 2010 relatives AT médecine AT surveillance a pour objet de permettre un professionnel médical d'interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical du patient, donc il nous semble satisfait une demande de retrait, celui de la Commission, c'est la nuit favorable sur le 354, l'article a précisé que le cahier des charges relatif aux expérimentations et surveillance dans le domaine de l'insuffisance rénale chronique intègre la dialyse à domicile, on a eu le débat hier sur le problème, l'insuffisance rénale chronique, donc c'est vrai que l'expérimentation des surveillance doit s'articuler avec celles par ailleurs engager son parcours de soins de ses patients, mais sur le fond, il a, par la commission qui n'appartenait pas à la loi de fixer les modalités de ces expérimentations, toutefois, nous avons souhaité avoir des éclairages de votre part Madame le Ministre, sur la place de la dialyse à domicile au sein des programmes engagés donc une demande d'avis du gouvernement, elle 36 rédactionnel, c'était un vif. à vous, Madame la Ministre, pour l'avis du gouvernement sur ces 4 amendements. concernant l'amendement 231 nous y sommes défavorables, parce que la télé-surveillance est un acte. Beaucoup plus complexe que la TV consultation consultation que la télé-expertise fait souvent appel à des dispositifs médicaux qui doivent montrer le service médical rendu autour de ces organisations et autour de ces dispositifs donc nous souhaitons poursuivre le cadre des expérimentations avec. Duel est terminé, je vous rappelle qu'un rapport au Parlement est prévu à mi-parcours, en juin 2019 mais clairement, la télé futur veillant s'ne nous paraît pas encore mûr, comédien Madame, de Roche pour rentrer dans le droit commun, nous avons impérativement à veiller à ce qu'elle apporte un service aux malades et qu'elle n'est pas potentiellement délétères donc défavorable pour cet amendement pour l'amendement de 366 pardon, nous nous considérons que cet amendement est déjà couvert puisque il est réalisable dans le cas des expérimentations de télésurveillance donc ces retraits sinon défavorable sur l'amendement 121 de la Commission, nous nous sommes tout à fait d'accord pour couvrir l'enfant l'ensemble du Champ de l'offre de soin et le secteur médico-social, donc favorable à votre amendement concernant le 354 rectificatif sur la dialyse à domicile, nous partageons votre intérêt pour les modes de prise en charge à domicile évidemment pour autant, la définition du périmètre des cahiers des charges relatif à la télésurveillance ne relève pas du domaine de la loi, aujourd'hui il n'y a pas d'expérimentation en cours, mais en revanche évidemment l'idée très intéressante, et elle pourrait être intégrée dans des expérimentations nouvelles nous allons-y travailler enfin l'amendement rédactionnel favorable. Donc passer aux amendements un par un, 231 il y a-t-il des explications de vote Monsieur Morisset. Oui, compte tenu des précisions apportées par Madame le rapporteur et puis d'engagement de Madame la ministre, d'attendre 2019 pour le rapport intermédiaire d'évaluation, je retire l'amendement. Retirer ensuite, explications de vote sur 366 rectifier bis : il est retiré. Retirez merci madame de roche, amendement 121 rectifier oui de la commission bien sûr hé oui du gouvernement. Qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, il est adopté, ensuite le 354 rectifier terre. Défendu par Monsieur Daudigny, la Commission a demandé un avis du gouvernement, le gouvernement a dit non

donc cette dimension de la dialyse à domicile dans les expérimentations de télésurveillance, hein, c'est plus restrictif que ce qui a été évoquée hier je retire l'amendement. Il a aussi retiré et puis l'amendement de précision rédactionnelle avec avis favorable du gouvernement numéro 122 qui et pour qui et contre qui s'abstient, il était adopté, nous passons à l'amendement 479 Madame Cohen, vous avez la parole. S'il y a eu, il y a un fort Monsieur le président, Monsieur le Président, la ministre, chers collègues, notre amendement visant à encadrer la pratique de la télé-médecine, avec l'élaboration d'une charte des bonnes pratiques de la télémédecine qui serait rédigé en concertation avec les professionnels de santé les de santé des établissements de santé etc, sur le latin médecine puisque nous en avons beaucoup parlé, nous aimerions 2 observations, une technique et l'autre éthique, la première technique c'est que il faut pas s'imaginer que la télémédecine, va, va, permet de trouver une solution aux déserts médicaux, puisque malheureusement dans nos campagnes, c'est le Corrézien d'origine qui parle très souvent, les déserts médicaux sont aussi des déserts numériques et que malheureusement pour cette forme de médecine, il y a des contingences techniques qui sont extrêmement exigeante et aujourd'hui pas satisfaites, voilà l'autre point plutôt éthique, c'est qu'il faudrait éviter de déshumaniser la médecine le praticien n'est pas un garagiste qui change des organes, c'est aussi un accoucheur des esprits et nous avons besoin de maintenir ce contact humain entre le praticien et son patient pour cette raison, nous souhaiterions vivement que nous puissions accompagner la réflexion auquel vous êtes engagé auprès de nos collègues du groupe GDR à l'Assemblée nationale pour mettre au point une charte de bonnes pratiques, merci. Votre avis madame la rapporteure. mais Madame la ministre, indiqué que la Haute autorité de santé sera également consultés sur les bonnes pratiques de télémédecine et donc un corpus de règles qui va se constituer et il ne nous a pas semblé utile de prévoir dans la loi une telle charte quel que soit son intérêt, nous faisons confiance aux professionnels pour s'organiser, c'est donc un avis défavorable.

bien sûr sur le désert numérique, nous avons le même constat que vous êtes que nous avons une urgence à travailler cette désertification numérique et c'est d'ailleurs une des priorités du secrétaire d'État au Numérique Mounir Mahjoubi que de couvrir ces territoires, de façon justement à pouvoir déployer notamment. Mais pas que la télémédecine concernant l'amendement proposé en fait, le code de la santé publique prévoit déjà que les acteurs d'un projet de télémédecine signent une convention entre qui organisent leurs relations et les conditions dans lesquelles ils mettent en avant des obligations qu'il incombe je pense que c'est déjà couvert mais au-delà de ça, je suis absolument convaincu comme vous que la télémédecine, ne peut pas remplacer la relation singulière médecin-malade, le fait qu'on examine un patient, bien entendu, c'est la raison pour laquelle j'ai saisi la Haute autorité de santé de façon à ce qu'elle nous aide à réfléchir à l'encadrement par exemple à identifier des symptômes ou des problèmes qui ne pourrait pas faire l'objet de télémédecine, je pense notamment à quelqu'un qui aurait très mal au ventre, nous savons tous, en tout cas les médecins qui sont dans la salle, qu'il faut poser une main sur le ventre et que ça ne peut pas se traduire par une téléconsultation, donc je pense que nous avons besoin évidemment de travailler collectivement, c'est la raison pour laquelle la Haute autorité de santé sera saisi une bonne définition des bonnes pratiques pour accompagner ce virage de la télémédecine, je pense, donc votre amendement est largement couvert par les orientations du gouvernement, il propose un retrait.

Qui est contre. Qui s'abstient, l'article 36 est adopté, nous passerons à l'article additionnel après l'article 36. Et à vous la parole monsieur Vatrin. Oui pour l'amendement 480 un autre amendement vise à limiter les dépassements d'honoraires en remplacement, en remplaçant le et mesures de la loi par un plafond défini par décret la négociation sur l'avenant numéro 8 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie était en en effet encadrer la maîtrise des dépassements d'honoraires, les signataires de la convention devait s'engager à maintenir ou à développer leur part d'activité en tarifs opposables constatées lors de la signature du contrat, mais c'est une contrainte de faible portée pour les praticiens qui avait une part réduite de leur activité déjà en secteur 1 cette contrainte leur procure d'ailleurs des avantages importants prise en charge de cotisations sociales sur les honoraires correspondants l'activité réalisée au tarif opposable et bénéfices des revalorisations des tarifs des remboursables applicable aux médecins exerçant en secteur 1 la mise en 9 de ce désir positif, a démontré ligne efficacité de cette contractualisation, j'en veux pour preuve le rapport d'activité 2016 de la direction de la conciliation de l'assurance maladie, qui a révélé que les refus ou les problèmes d'accès aux soins ont progressé de 8 pourcent entre 2013 et 2016 et le motif le plus signalé celui du refus de tiers payant pas les dépassements d'honoraires, nous vous proposons donc d'encadrer réellement la pratique des dépassements d'honoraires en fixant un plafond maximal par arrêté. Merci l'avis de la commission Madame la rapporteure. Alors, il nous a semblé que la notion actuelle de tact et mesure, et moins rigide qu'un plafond uniforme qui sera fixé par décret, elle permet de prendre, donc on a diversité des situations tout en protégeant les assurés, c'est donc une demande de retrait où un avait déjà. Bien, Madame la Ministre votre avis. la convention médicale de 2000 16 heures. Prévu une option pratique tarifaire maîtrisée Octomom avec une déclinaison spécifique pour les chirurgiens, les obstétriciens afin d'attirer de nouveaux adhérents à ces contrats d'accès aux soins et les conditions d'adhésion et tarification allochtones, se sont assouplies à plusieurs égards cet accord, il commence à porter ses fruits, entre avril et août 2016, la tendance à l'adhésion des nouveaux médecins assez pratique est en hausse, avec près de 10000 médecins qui ont adhéré à l'aube. Tom et adopta me chirurgie obstétrique, donc il nous paraît que ce dispositif de régulation est en train de trouver sa place, que les médecins adhère de plus en plus facilement et ne nous paraît pas opportun d'y mettre fin et de revenir sur les accords signés qui pourrait provoquer des déconventionnement donc nous vous proposons un retrait avec ces éléments et sinon avis défavorable. Il est maintenu, donc avec 2 demandes de retrait et avis défavorable, donc de la Commission et du gouvernement. Et pour qui est con. Qui s'abstient l'amendement n'est pas adopté article additionnel après l'article 36 Madame Cohen, vous avez la parole. est quand même un amendement de repli puisque nous sommes opposés à toute barrière financière aux soins dépassements d'honoraires, franchises médicales et participations forfaitaires de de tous genres, donc cette fois-ci, nous pensons qu'il serait nécessaire de rétablir les sanctions financières. Qui ont été supprimées par la loi HPST alors vous nous dites, Madame la Ministre, énoncé même rapporteur excusez-moi tact et mesure, c'est c'est mieux adaptés, moi je vous donne un exemple concret vécu il y a 2 jours, dans le quartier dans lequel se situe le Sénat 5 minutes de consultation chez chez un ophtalmo 150 euros, je ne sais pas s'il s'agit de tact et mesure, mais on n'a pas la même conception des choses, donc voilà, on est dans les dépassements d'honoraires. Plus plus plus, alors, et moi je le dis sur une expérience concrète mais dans son rapport sur la sécurité sociale, la Cour des comptes a jugé inefficaces les mesures qui sont mises en place et qui ont été rappelés par Madame la Ministre, pour lutter contre les dépassements d'honoraires en 10 ans la proportion du nombre de spécialités installés en secteur 2 a augmenté, passant de 39,2 pourcent au total des spécialistes libéraux en 2006 à 44,3 en 2015 pour quelques spécialités les dépassements sont presque devenus la norme 84 pourcent des gynécologues en pratique 69 pourcent des ophtalmologues offres ophtalmologiste nous sommes cette fois-ci, d'accord, donc avec la Cour des comptes qui a jugé les effets très limité pour un coût très élevé car si la hausse du taux moyen des dépassements a bien été enrayée, passant de 55 pourcent 2011 à 51 en 2015 c'est au prix d'une forte dépense publique puisque, pour éviter un Euro de dépassement, l'assurance maladie a ainsi dépensé 10 euros, la cour a pas ailleurs d'appareils hors dénoncer la tolérance des Caisses d'assureurs maladie à l'égard des gros, des passeurs, peut-être que l'exemple que je vous ai donné fait fait partie d'ailleurs des gros, des passeurs avec seulement 1400 sanctions prononcées entre 2012 et fin 2015 à l'égard des médecins refusant d'infléchir leur pratiques tarifaires, c'est pour ces raisons que nous proposons de rétablir cette sanction pour les professionnels de santé qui ne respecteraient pas cet article, ainsi d'ailleurs que ceux qui pratiquent des refus de soins. Merci madame la rapporteure votre avis. sur l'amendement 480 il existe déjà des sanctions pécuniaires contre des professionnels de santé, dans le cas de dépassements d'honoraires abusifs, la section des assurances sociales, de la Chambre disciplinaire a par ailleurs compétente pour connaître des photos des abus, occasion de soins dispensés aux assurés, il n'a pas semblé opportun à la commission d'ajouter un nouvel étage à cet arsenal de sanctions, c'est donc une demande de retrait ou un avis défavorable. Madame la ministre avait du gouvernement. Oui, pour les mêmes raisons avis défavorable. Madame Cohen, vous avez la parole. J'ai pas la prendre très longtemps, mais je ne vois pas en quoi, on peut penser que ces mesures mises en place sont efficaces. Donc, la Cour des comptes quand même dit il y a eu entre 2012 et 2015 14 sanction donc ça veut dire qu'on laisse courir. Donc. Il est maintenu, on va consulter notre assemblée amendement 480 avis défavorable de la commission avis défavorable du gouvernement qui est pour. Ces contrats. Qui s'abstient, il n'est pas adoptée après l'article 36.

J'ai eu l'honneur de de participer à la rédaction de la loi HPST inscrire dans le marbre la télémédecine et la télé rare qui est une véritable avancée scientifique et technologique, et qui permet aux territoires les plus vrai que reculer d'avoir accès à un radiologue main mais malheureusement la législation actuelle sur la télémédecine ne permet pas de garantir que les actes de télé radiologie soit réalisée conformément à la réglementation, je m'explique : nous voyons apparaître des saucisses low-cost qui interprète des scanners qui sont situées au Diable Vauvert. Sur lequel on a aucune action sur la signature, on ne connaît pas le radiologue on ne sait pas s'il a des bon diplôme. Et ces sociétés locales ne garantissent pas le respect de la réglementation de la déontologie. Et là, je ne parlerai même pas des tarifs médicaux réglementaire, je m'abaisserait pas là, je ne parlerai simplement de qualité, un acte de radiologie comme un acte médical doit être un acte de qualité, donc il y a une rupture d'égalité entre le patient qui va aller dans le 6ème arrondissement, rue de Vaugirard, il va avoir un radiologue, avoir un scanners et celui qui habite. Dans le Châtillonnais, au nord de la Bourgogne, où il sera son scanners sera un peu un interprété par quelqu'un qui habite à Abou Dhabi, donc cet amendement permettra de définir des règles communes, comme par exemple celles inscrites dans la charte de la de télé radiologie élaboré par le Conseil de professionnels de la radiologie et cosignée par le Conseil national de l'Ordre des médecins et de telles règles. sont des règles qui permettent de garantir le respect des conditions d'un acte médical pour le patient de cet art édification et du traitement des dossiers des parents

Monsieur le Président, Madame la ministre de pas être très long parce que l'amendement est identique à celui de notre collègue, il l'a très bien expliqué donc je partage entièrement cette position, donc c'est pour ça, je soutiens l'amendement. Très bien amendements identiques encore le 324 Monsieur Daudigny. Oui, Monsieur le Président, Madame le Ministre, mais chers collègues même amendement argumentation présentée par votre collègue monsieur Pères était excellente, je la partage vraiment insister sur cette idée que, avec le développement de nouvelles pratiques utilisant des technologies modernes nous prenions garde à l'installation, nombre de sociétés low-cost qui est venu hier et cela a été fort bien dit, à la qualité des travaux médicaux qui pourraient être rendus

alors le le conseil départemental Bien décidé un projet magnifique fibre à la maison pour 2020 avec la règle, l'État, la région, le département et les communautés de communes, donc la médecine va pouvoir se réaliser aussi encore. Merci Merci l'avis de la Commission sur ces 4 amendements identiques. les inquiétudes soulevées par nos collègues bien défendu par Alain Houpert sont sont sont fortes parmi les professionnels de de santé mais aussi parmi parmi les patients et et et la Commission a souhaité demander l'avis du gouvernement. D'accord sur ces quatre identique, hé bien l'avis du gouvernement Madame la milice. Oui, Monsieur le Président, je suis totalement en accord avec le constat que vous faites et je suis moi-même sidéré de voir comment certains établissements contournant fait se sont gouffre dans un vide juridique ou contourner le code de la santé publique pour effectivement adressé tels ou tels clichés parfois dans d'autres pays avec une qualité d'interprétation qui est questionnable, donc c'est un sujet dont je m'étais déjà emparé lorsque j'étais un total autorité de santé que je souhaite évidemment très bien encadré, aujourd'hui il me semble cependant que ce que nous allons mettre en place pour la télémédecine, médecine et la télé-expertise, là on est dans le cas de la télé-expertise en puisque ce sont des clichés adressé à un médecin, donc c'est vraiment le cadre réglementaire qui va être discutée dans la convention médicale et qui va permettre d'une part, de négocier les tarifs d'autre part de négocier les conditions, donc je pense que, avec l'entrée de la télé-expertise dans le droit commun, nous allons permettent de cadrer correctement ces pratiques déviantes, nous en sommes absolument tous conscients, c'est vraiment l'objectif de cette convention, qui est de cette négociation qui débute je rajoute d'ailleurs que je saisis la Haute autorité de santé pour encadrer encore mieux certains actes et d'avoir un guide des bonnes pratiques qui soient adossés à certains actes, je pense que nous sommes en train de faire le travail de régulation nécessaire, je ne pense pas que votre amendement telle qu'il est rédigé, qui dit : la définition des actes de télé radiologie ainsi que leurs conditions de mise en oeuvre et de prise en charge financière seront fixées par décret chance quoi que ce soit ce que nous proposons, en fait, la la télé radiologie s'étant en fait complètement daté d'expertise, ce n'est rien d'autre, donc ça rentre, ça rentre dans le droit commun et ça va être négocié dans la convention médicale vous proposait de fixer par décret, mais voilà la la convention vise justement à définir le cadre et à réguler les tarifs, moi je pense que votre amendement va être couvert par l'action du gouvernement, je peux m'engager devant vous, avoir une attention toute particulière à la mise en oeuvre de cette convention médicale dans le Champ de la télé-expertise en en télé radiologie mais il me semble que nous sommes en train d'organiser ce Champ d'expertise vous propose un retrait sinon défavorable mais je tenais à vous faire part de mon âge de mon engagement personnel sur ce sujet. Monsieur. Madame la Ministre, vous dites que la réalité, la radiologie et de la. De l'expertise, pour moi c'est un voeu pieux parce que, en tant que radiologue je constate chaque jour, des erreurs de diagnostic et quelquefois un diagnostic qui ne correspond pas aux patients, donc là il y a un problème on on exige de la traçabilité pour les aliments

des compétences, nous avons des radiologues qui sont dans les hôpitaux qui sont en retraite qui ne demanderaient qu'une chose, continuer, continuer à exercer, continuer à aider leurs patients, parce que la médecine, c'est une mission, c'est une vocation n'est-ce pas mon cher collègue, 1 1000000, c'est quelque chose qui nous habite, voilà, donc je ne suis pas d'accord avec vous un administré, rassurons les radiologues et ceux qui font de la télé radiologie, ce sont des radiologues qui sont pratiquement en secteur 1, rassurons les radiologues et rassurant et apportons de la qualité aux patients merci. Monsieur le président de la commission. Merci Monsieur Président je je vais évidemment soutenir l'action d'Alain Perrin sur le sujet de la télé radiologie mais je voudrais aller au-delà parce que nous assistons actuellement Madame unissez si vous en êtes consciente à un véritable dévoiement de l'acte médical,

votre médecin ou fait une consultation ou enfin, il y a eu hostiles ou fait une prescription et bon ben certains organismes complémentaires vous au cas où votre médecin se tromperaient consultez notre propre médecin par téléphone qui vous dira s'il a raison ou pas, je veux dire clairement on est actuellement en période d'urgence parce que le numérique prend le dessus sur l'acte médical et humain, mais je crois que vraiment je soutiens à fond l'acte, pardon, l'amendement de d'Alain Houpert et je dois dire, madame la ministre, il faut qu'il y a urgence dans des vraiment d'actualité Madame Goulet, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, même le milieu, je vais aussi soutenir cet amendement, moi je ne suis pas ni médecin ni ni radiologue mais je suis un malade en puissance et libéralisation

je voudrais profiter de du temps qui me restait même pas d'ailleurs pour dire à la upper qui se qui se rassure sur la qualité des soins Abou-Dhabi, je préside le groupe des pays du Golfe, et je voudrais vous dire que la qualité des soins ou débit est parfait, donc fera peut-être leur du procès-verbal, merci. Bien, donc, madame la ministre, à nouveau saisi. Oui, Monsieur le Président peut peut-être juste expliquer ma position d'abord je ne souhaite pas du Berry, stations de la médecine clairement pas et et pas plus de radiologie que n'importe quel autre acte, je pense que vous avez compris maintenant, comment je me positionne pour la qualité des soins, pour autant, je pense qu'il y a aujourd'hui des pertes de chance dans certains territoires, je pense, notamment, des territoires, sur lequel on pourrait tout à fait avoir une IRM qui fonctionnent la nuit pour avoir un diagnostic sur un accident vasculaire cérébral, sans qu'il y a des radiologues présents parce que nous savons que nous avons du mal et les avoirs et vous savez très bien qu'un acte de trop bec Tommy par exemple va dépendre d'une IRM et le transport du malade en urgence va dépendre de l'IRM, je pense que il faut qu'on arrive à développer ce type de télé-expertise à distance pour sauver certains hôpitaux de proximité et permettent, parce qu'on parlait beaucoup de déserts médicaux et d'accès aux soins, la typiquement c'est permettent l'accès aux soins de proximité tout en n'ayant pas un radiologue de garde la nuit pour être à côté de l'IRM, donc je pense qu'il y a des sujets sur lequel ça sera un vrai service rendu au patient, ça veut pas dire qu'il faille Hubert la radiologie française c'est vraiment pas l'objectif, donc c'est pour ça que je souhaite encadrer que la la Haute autorité de santé explique bien le type d'actes qui doivent bénéficier telle expertise et ceux qui ne le doivent pas, ou moins, il faut qu'un médecin, par exemple, je pense, quand on fait une même mot, il vaut mieux que le médecin a examiné 5 de la femme, on ne sait bien et donc il y a des actes ou il faut que le médecin soit présent examine et d'autres ou, au contraire, nous savons très bien que la télé-expertise à distance va rendre un service aux malades, donc tout ça mais vient d'être organisé sur le territoire, c'est ce que nous allons faire et la raison pour laquelle je ne suis pas favorable à votre amendement c'est c'est vous proposer que la prise en charge financière de ces actes de télé radiologie soit fixée par décret, ce serait le seul acte médical dont le tarif serait fixé par décret, ça ne paraît pas judicieux et donc je maintiens mon avis défavorable, je voulais donner cette explication merci. Donc, nous allons passer au vote dès 4 amendements identiques avec. La Commission avait demandé l'avis du gouvernement, finalement vous dites oui ou non. je, je dis oui sur le sur l'objectif mais je partage l'avis de la ministre quant à la rédaction et notamment à ce que la fixation par décret qui qui qui souhaite la négociation conventionnelle, sur le fond, pas. Tâche tous cette volonté qu'en effet il y a pas une marchandisation de la télé-expertise et que mais mais l'exemple qu'a donné, madame la ministre sur les AVC sur l'exigent la possibilité d'accélérer la trompe le délai pour la trompette, mais quelque chose qu'on vit dans tous nos territoires, donc la rédaction de l'amendement en fait quand même du du juridique et des législatives et et pour ma part, moi je, alors le président est favorable, la rapporteure n'y est pas, donc c'est sagesse. Donc sagesse de la Commission. Avec rapporteur qui est contre le rejet et contre du gouvernement. Qui est pour.

nous passons après l'article 36 l'amendement 482 c'est Madame Cohen non Monsieur Oizo, il y a. Oui, raté, monsieur le président, un ministre mais, chers collègues, nous avons été interpellé au sujet de la situation des praticiens à diplôme hors de l'Union européenne qui exercent dans les hôpitaux français sur des contrats précaires de courte durée, sans perspectives d'évolution ni de stabilité dans leur carrière et pour des rémunérations souvent inférieures à celle de leurs confrères du 1er en France ou dans l'Union européenne, ils forment en quelque sorte la masse des travailleurs détachés de la médecine détenteurs de diplômes post-doctorants en France mais la procédure d'exercice ne prend pas en considération leur expérience en France et le nombre de postes ouverts aux candidats non résidents est quasi nul, les besoins praticiens médicaux en France, nous l'avons dit je le répète et les inégalités d'accès aux soins dans les déserts médicaux, médicaux sont grandissants, en permettant l'exercice aux praticiens recrutés dans les établissements de santé avant le 31 décembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2024 notre assemblée apporterait une vraie amélioration à ces problèmes, nous proposons pour ces raisons de reconduire les épreuves de vérification des connaissances pour les praticiens, dès lors qu'il justifie d'au moins 2 mois d'exercice, entre le 31 2016 et la date de publication et d'avoir exercé 3 ans en équivalent temps plein la disparité des statuts des praticiens et les inégalités qu'elles entraînent, ne sont plus acceptables d'autant, que nous sommes face à des professionnels de santé diplômés qui disposent de diplômes et qualifications équivalentes à leurs homologues professionnels nationaux à responsabilités égales, les praticiens doivent avoir une rémunération similaires ce n'est pas en continuant de recruter en contractuels, les professionnels de santé hors Union européenne que nous améliorerons le service public rendu, ils ne sont pas destinés à demeurer la variable d'ajustement de planning, notamment le soir et le week-end et dans les services d'urgence télé le sens Madame la Ministre de notre amendement merci. Merci madame la rapporteure, l'avis de la commission. Alors, l'enjeu est d'accompagner les professionnels concernés, tout en demeurant bien évidemment exigeant sur la qualité des soins, il nous a semblé que cet amendement rendrait pas forcément dans le cas du du PLFSS et peu. Peut-être prématuré d'engager une évolution sur le sujet, néanmoins ne souhaite tuant, Madame la Ministre que que vous puissiez apporter des garanties sur sujet des des praticiens et obtenu un diplôme hors Union européenne et donc la Commission souhaite avoir l'avis du gouvernement. Madame la Ministre votre avis. Monsieur Président oui c'était un un sujet sur lequel nous sommes en train de nous pencher, il s'agit d'État du des des praticiens diplômés hors état de l'Union européenne et vous proposez en fait de poursuivre par votre amendement leur activité jusqu'au 31 décembre 2024. Or il se trouve que je travaille sur ce sujet, je souhaite améliorer en 2018, la procédure d'autorisation d'exercice pour l'ensemble de ces praticiens et et plutôt que de se limiter part votre amendement a simplement reconduire une nouvelle fois un dispositif transitoire à l'identique du précédent et réservé à une catégorie spécifique de preuves je suis en train de concevoir une procédure qui prend appui sur les acquis du 3ème cycle des études médicales qui vient d'être rénové et sur lequel je vais engager ces praticiens de façon à ce qu'il aient soit une validation des acquis de l'expérience soit accès en tous les cas à une pratique qui ne soit pas simplement dérogatoire de ce type, je vous propose de retirer votre amendement sinon j'y suis défavorable. Votre proposition va plus loin que ce que nous demandons donc nous retirons notre amendement merci.

la commission de hiérarchisation des actes et prestations à, de par la loi pour mission d'établir les règles, il y a ation des actes de sa profession et de valider cette hiérarchisation qui en résultent actuellement concernant la détermination du coût de la pratique affectés à chaque acte, l'article R-162 52 du code de la Sécurité sociale, indique que l'une canne défini le thème de l'acte ou de l'appréciation dans le respect des règles de hiérarchisation levier de cet amendement est de permettre à la commission de il y Hargeisa Sion des actes et prestations qui est une instance paritaire de piloter et de déterminer la procédure d'évaluation du coût de la pratique des actes. Merci l'avis de la commission. détermination d'Éric dévaluation du tarif associé à chacun ou pour déterminer son préalable, à savoir le coût qui serait associé à pratique si c'est le 2ème cas ça sans que la demande est satisfaite par la pratique des mais en tout état de cause, compte tenu de l'imprécision de la rédaction, il nous a paru difficile d'intégrer cette modification, c'est donc un avis défavorable. Madame la ministre à vie du gouvernement. Oui, monsieur le président de la commission de hiérarchisation des actes et prestations aujourd'hui elle mobilise des experts pour apprécier le niveau en fait de mobilisation d'un professionnel en fonction de la complexité de cette expertise est reconnue font tout le dispositif d'inscription il y a incitation des actes, c'est en revanche, l'assurance maladie de procéder à l'inscription à la tarification de la pratique à partir de cette hiérarchisation, donc si on étendait les compétences des chapeaux de la pratique, cela reviendrait à bouleverser les règles de fixation des tarifs par l'assurance maladie en transformant des experts scientifiques en analyste économique, donc nous sommes défavorables à cet amendement. Merci madame la ministre. Monsieur retire donc maintenant un amendement de la commission Madame Desroches Oui alors cet amendement fait tant à rétablir la procédure d'inscription accélérée des actes la nomenclature qui était dans le texte initial du gouvernement et qui a été supprimée par l'Assemblée nationale et cette procédure passe par un dessaisissement temporaire des chapeaux en quatre blocage alors le choix de la solution, nous préconisons et résulte d'une volonté de conciliation 2 objectifs, c'est l'association des partenaires conventionnels doit toujours être privilégiée lorsqu'il s'agit de faire évoluer les cadres et conditions d'exercice professionnel, l'accès des patients l'innovation thérapeutique doit cependant constituer une priorité et de ce point de vue, le dispositif proposé par présent article apparaît relativement équilibrée, il convient en 1er lieu de souligner que la rédaction proposée reconnaît une simple faculté d'intervention à et ne lui donne pas obligation d'intervenir à l'issue du délai prévu pour la prise de décision des chats et en sort le dispositif proposé préserve la compétence de principe de Chaplin deviendront pas de simples instance consultative ses 6 mois leur dessaisissement ne sera que temporaire, la rédaction proposée pour l'article prévoyant impossibilité d'une nouvelle inscription suivant la procédure de droit commun, l'échappée auront d'ailleurs la possibilité lors de ce nouvel examen de voter une hiérarchisation différente de celle établie par une enfin le délai proposé pour la phase de hiérarchisation 11 mois au maximum paraît raisonnable, on peut imaginer qu'une scission éclairé puisse survenir dans ce délai, au total, l'application de l'ensemble de la procédure aboutira n'inscription d'un acte nouveau, à un an et demi, ce qui peut apparaître comme un maximum déraisonnable qu'on a connu des délais beaucoup plus longs, néanmoins pour répondre en effet à ce que pouvaient des interrogations des chapes

ou scientifiques particulière, donc nous nous préférions la rédaction initiale de l'article plutôt que celle votée à l'Assemblée nationale avec cette souplesse qu'on a mis sur la progression enquête difficulté c'est donc l'objet de cet amendement. Il y a un l'avis du gouvernement Madame la milice. Monsieur Président, peut-être par souci de cohérence, nous avions donné un avis favorable à l'amendement proposé par le rapporteur à l'Assemblée nationale et donc on va rester fidèle à à cet accord qu'on leur a donné donc défavorable aux vôtres, non je ne préfère personne Monsieur. y a pas d'explication de vote, donc nous allons passer au vote de cet amendement avis favorable de la commission avis défavorable du gouvernement qui est pour. Ces contrats. Qui s'abstient c'est un amendement qui était adopté je j'informe notre assemblée. Qu'il est midi et que nous allons aller jusqu'à 13 heures pour lever la séance de ce matin. Voilà 338 rectifier Monsieur Jomier. Merci monsieur le président, cet amendement qui relatifs au protocole de coopérative coopération pardon vise à répondre à une difficulté qui minore le recours à ces protocoles de coopération sa difficulté étant des télés important de d'instruction et de réponse et on constate que dans un certain nombre de cas significatif, ces délais sont induits par une difficulté à apprécier la pertinence du protocole au regard des priorités nationales, et donc l'amendement que je vous propose, vise à mieux préciser ses priorités nationales afin de d'accroître le recours au protocole de coopération qui sont nécessaires. Merci l'avis de la commission. Alors je partage bien évidemment la préoccupation exprimée par les auteurs de l'amendement d'ailleurs, ça paraît très difficile de ne pas la partager tant la formulation retenue et là, cependant, pour la même raison, nous sommes ta précision inutile le domaine visé est si vaste que je ne vois pas comment les priorités retenues, pourrait ne pas y correspondre, donc il y a en plus un problème de rédaction, mais ça c'est un peu ce qu'on a, donc c'est une demande de retrait ou un avis de façon. Madame la Ministre votre avis. Monsieur le Président, je je remercie, Monsieur le Sénateur, je mets de de veiller à ce que ma stratégie nationale de santé actes axes prioritaires, inscrit dans la loi, mais de fait, en fait, nous travaillons à un arrêté pour fixer les priorités pour les protocoles de coopération donc en fait nous allons couvert via un arrière un arrêté et donc je vous propose un retrait. Monsieur Jomier, que répondez-vous oui vous retirer. Donc maintenant demande coordination 124 Madame rapporteur coordination avis du gouvernement, sur cet amendement de coordination. Favorable merci. Donc, avis favorable au gouvernement. Et qui est pour. qui est contre. S'abstient, il est adopté, nous allons passer au vote de l'article 37 dans son ensemble qui est pour. Qui et contre qui s'abstient, il était adopté, nous poursuivons après l'article 37 le 191 rectifier bis madame Moret. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, le code général des collectivités territoriales à son article de 2223 42 dispose que seul un mais de cinq peut délivrer un certificat attestant le décès et autorisant de ce fait, la fermeture du cercueil, ce document officiel permet d'établir que le décès ne suscite pas d'interrogations d'ordre médico-légal et que le défunt n'est pas mort d'une maladie contagieuse répertoriés par l'Organisation mondiale de la santé, charge de la prise en charge par l'époque funèbre l'imprimé correspondant et rempli partout mais de inscrit à l'ordre des médecins sur la base du volontariat, l'établissement des certificats d'essai a été abordée dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2016, celle-ci a prévu une prise en charge forfaitaire, décès, certificat établi au domicile parler mais de 5 dans le cadre de la permanence des soignants, les textes d'application ont été publiés le 10 mai 2017 pour autant le problème récurrent du manque de praticiens médicaux pour dresser le constat de décès n'a pas été réglés en effet, il devient très difficile, notamment dans certaines zones que mais de 5 se déplace dans un délai raisonnable, ce qui n'est pas acceptable du point de vue administratif ni sur le plan humain en laissant au seul mais de c'est la possibilité de délivrer un certificat de décès, la loi ne tient pas suffisamment compte de l'évolution de notre société et du développement des déserts médicaux, c'est pourquoi il est souhaitable de prévoir un dispositif plus souple pour tenir compte de ce phénomène qui touche désormais les espaces ruraux, mais aussi certaines villes, telle est l'objet du présent amendement en en maintenant qui permet s'espérant de règles adoptées au Canada par le Canada que le certificat de décès puisse être établi par l'infirmière ou les fermiers et il y a en dispenser des soins durant la dernière maladie lorsque l'issue de celle-ci était prévisible. Oui, avis de la commission. Cet amendement a suscité un un grand débat en commission, certains étant favorables. Mais gare aux difficultés qu'a souligné, notre collègue Maurer et chaussures, parfois les difficultés à voir un médecin pour établir et sur le cadre Kelly mais qui est celui que ça puisse être établi par l'infirmière, l'infirmière qui a dispensé les les soins lors de la maladie lorsque l'issue fatale était prévisible, néanmoins, on est sûr du médico-légal il y avait aussi des oppositions fortes par rapport à cela au sein de la commission et et des risques posés de ce qui est quand même l'engagement de signature d'un certificat décès notamment ce qu'il faut dire qu'il y a pas de de morts suspectes, donc, donc, en fait, et puis la notion de prévisibilité du décès sur plan législatif est assez, assez complexe à définir donc la Commission souhaitait avoir l'avis du gouvernement. Eh bien, Madame la Ministre votre avis. Oui, Monsieur le Président Madame la rapporteure, vous avez raison, c'est un amendement qui est intéressant parce que vous soulevez une vraie question : une vraie problématique de Téhéran, je ne suis pas sûr que la façon dont s'est rédigé et de l'inscrire dans lequel législatives va nous aider à régler le sujet en fait, je pense qu'il faut effectivement travailler avec le ministère de l'Intérieur, c'est un acte médico-légales que nous devons travailler également en terme de délégations de tâches sur l'encadrement, je ne pense que l'amendement telle qu'il est rédigé nous poserait pas mal de problèmes de mise en oeuvre, donc je vous propose d'y travailler de revenir vers vous, peut-être pour le prochain PLFSS mais peut-être que ça ne sera pas du domaine législatif, mais certainement, nous allons explorer la la piste que vous proposez, je vous propose un retrait sinon défavorable. Vous répondez quoi madame. Au vu des des avis du de apporterait de madame la ministre, et au vu de de l'engagement qui est pris donc pour travailler sur cette question qui me paraît très importante pour nos territoires en matière de simplification, je retire l'amendement. Retirez donc nous passons à l'article 38 avec 2 amendements faisant l'objet d'une discussion commune : l'amendement 325 Monsieur Daudigny, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président Madame la milice mais, chers collègues, faire une présentation rapide de cet amendement 325 qui concerne l'activité de rétrocession assis mais essentiellement par les établissements publics de santé cet article 38 introduit une possibilité de variations et de réduction de la marge dans ce sens Saadat réduction en fonction du prix de cession de la spécialité pharmaceutique l'idée peut paraître cohérente de bon sens, la crainte est que cette baisse des marchés et donc de la recette globale remettent en cause l'activité de rétrocession la proposition d'amendement, disons que dans ce domaine, a gardé le monde ancien, et à restaurer une marge fixe pour les établissements de santé, je vous remercie. la marge des médicaments de la liste rétrocession est fixé de manière forfaitaire et et non par un pourcentage reposant sur prix du médicament, elle, actuellement fixé à 22 euros par un arrêté 2009 et c'est vrai qu'il ne paraît pas absurde pouvoir diminuer ce montant forfaitaire lorsque les produits sont peu coûteux, madame le Ministre pourra cependant nous apporter des éclaircissements sur l'interprétation qui sera retenu contre au terme de compte tenu de la modicité du prix de cession de la spécialité, mais la Commission a fait une demande de retrait ou sinon un avis défavorable.

cette modulation sera effectuée selon le prix du médicament, la modulation de la marge en fonction du prix du médicament a déjà appliqué pour les médicaments vendus par les pharmacies d'officine sans que cela ne pose de difficulté sur la qualité de la distribution, il est donc difficile aujourd'hui de justifier le paiement par l'assurance maladie, d'une marge de 22 euros par exemple pour un médicament dont le prix ne serait que le 2 ou 3 euros et c'est pourtant la situation actuelle, il ne s'agit évidemment pas de remettre en cause la qualité du circuit de distribution dès midi. également dans les établissements, il s'agit simplement de mettre en cohérence le montant de la marge avec le prix du médicament pour les produits très peu chers, donc, nous vous proposons un retrait sinon défavorable. Bien donc. Retrait ou des feux Monsieur Denis. Maintenu donc y a un avis défavorable de la commission, un avis défavorable du gouvernement qui est pour.

c'est un amendement de manque Honegger Bruno Gilles, qui a pour objet de rappeler que la fixation unilatérale d'un tarif unifié la vocation à intervenir de manière subsidiaire, c'est-à-dire à défaut d'accord entre le comité économique des produits de santé et l'entreprise concernée. Avis de la commission madame la rapporteure. et nous sommes cependant que la modification proposée par l'amendement aboutira à vider de sa substance le mécanisme qui est proposée par l'article 38 qui vise justement, instituer pour les médicaments sucer rétrocéder un tarif unifié distinct du prix, l'idée est d'inciter les établissements de santé que les produits les moins chers, dans le cas du mécanisme de l'écart médicalement indemnisables je rappelle par ailleurs que le prix des médicaments distribués à l'hôpital et libre et fait l'objet d'une négociation entre les laboratoires établissements, c'est donc une demande de retrait ou un avis défavorable. Madame la ministre, la vie du gouvernement. il n'y a pas lieu de préciser que le tarif unifié relève du Champ conventionnel, ce serait contraire au principe même de la mesure qu'il ferait et ferait croire que ce tarif unifié constituerait une voie usuel de fixation des tarifs alors qu'il s'agit d'une solution pour surmonter un blocage, donc nous sommes défavorable à cet amendement. Karoutchi. Devant l'unité de la réponse, je pense que Bruno Gilles, ne m'en voudra pas, l'amendement est retirée

oui, c'est effectivement un amendement de mon collègue Bruno Gilles, qui a pour objet de garantir que les médicaments de même indication de même visée thérapeutique similaires en termes de composition qualitative et quantitative ne puisse pas tirer argument d'une protection de breveter pour contourner la possibilité de l'éventuelle application un tarif unifié selon les modalités prévues par cet article. Merci l'avis de la commission. nous avons souhaité avoir votre avis Madame la ministre pour sur la porte et l'objectif de la formulation qui est celle de l'article 38. Votre avis. Je suis embêté en fait par cet amendement parce que il est trop enfin non en fait je suis défavorable, pardonnez-moi, mais je vais vous expliquer pourquoi, non monsieur vous expliquer pourquoi, monsieur le sénateur, c'est parce qu'en pratique, vous avez des produits génériques qui peuvent être tout à fait similaire en termes de principes actifs, mais dont l'indication va légèrement varier parce que telle des laboratoires aura déposé une indication plus restreinte qu'un autre, et donc en fait, la façon dont l'amendement et rédigé va permettre énormément de contournement à la règle d'unification tarifaire, c'est une façon fait de détourner complètement l'article de son intérêt, j'ai plein de médicaments en tête, donc moi je vais pas vous les il mais mais je voulais voilà je vous déconseille tous d'aller dans cette voie-là parce que nous n'aurons plus moyen de réguler l'une les tarifs donc défavorable. Bien, monsieur Karoutchi. Bien fait de venir ce matin enfin devant la la la force de conviction je comme je veux pas rendent les gens plus malades qu'ils ne le sont, je retire l'amendement bien quelle sagesse monsieur Karoutchi donc nous passons au vote de l'ensemble de l'article 38 ce qui est pour. Qui et contre qui s'abstient, il était adopté, nous poursuivons la discussion après l'article 38 Madame Cohen monsieur battra.

La liste des critères n'est pas n'est-ce limitative 1 les éléments cités peuvent donc, le cas échéant et prend en compte par le dans sa négociation avec les laboratoires pharmaceutiques, il n'a pas paru utile de porter ces éléments dans le texte de loi, d'autant qu'il y a plusieurs problèmes de rédaction, c'est donc une demande de retrait ou un avis défavorable. bien, Madame la Ministre votre avis. Je suis défavorable à cet amendement, non pas que je ne m'intéresse pas aux critères de fixation du prix des médicaments mais je pense que c'est un un amendement qui est est une fausse bonne idée, d'abord, il a beaucoup d'obstacles juridiques parce que les informations. Sur le coût de fabrication relève du secret des affaires, elles sont en plus hors de portée du législateur français, l'industrie pharmaceutique est en en en général une industrie mondialisée, donc il serait totalement impossible de contrôler l'exactitude des déclarations des laboratoires. Et en plus je pense que ce qui compte le plus pour fixer le prix du médicament c'est le prix d'investissements de R&D du laboratoire puisque son prix de facture fabrication donc pour toutes ces raisons, je suis contre, secrétaire, bien que votre objectif je le partage. Merci, Madame Cohen, explications de vote. d'où notre amendement qui est tout à fait perfectible, mais c'est un un réel problème avec une complexité certaines donc nous entendons les, les, les arguments et, à cette étape de de d'autres réflexions, et compte tenu des des moyens limités qui sont offerts aux sénateurs et sénatrices que nous sommes sur le plan législatif puisque nous sommes toujours contraint avec la les articles 40 et 41 de limiter des fois nos propositions, je veux quand même attirer votre attention madame la Ministre sur quelque chose qui pourrait nous être utile au niveau des des de la problématique

en oeuvre la politique de l'AP-HP en matière d'équipements et de produits de santé : médicaments, dispositifs médicaux réactifs et consommables de laboratoire, équipements médicaux utilisés à l'AP-HP nous pensons que peut-être il serait utile de réfléchir ah au fait que cet établissement puisse élargir son son son Champ d'action au-delà de l'AP-HP, mais pour qu'il en soit ainsi, donc ça serait en quelque sorte un comment dirais-je une prémisse d'un d'un d'un pôle public du du du médicament donc un laboratoire public mais pour qu'il en soit ainsi, il faudrait l'aide de l'État, parce que c'est pas, c'est pas possible autrement, c'est-à-dire qu'il faut effectivement des moyens qui soient donnés tant humains que financiers, alors j'ai bien conscience que l'argent on va beaucoup plus loin que mais comme je sens depuis le début du débat que Madame la la ministre et est attentive aux propositions qu'on peut émettre je me raccroche à cette discussion pourrait éveiller toute son attention et lui dire qu'on est à sa disposition pour échanger Please à fond, merci. Donc vous maintenez votre amendement. Oui oui bien Donc l'avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il n'est pas adoptée après l'article 38, il y a un amendement 125 de la commission. Cet amendement est relatif aux athées urnes le débat lors des discussions générales et c'est vrai qu'on aurait souhaité, souhaité déposer des amendements, notamment par rapport à l'extension d'indication et la réduction des délais lorsqu'il y a une extension d'indication

détermination du montant remise au type de produits TU ainsi que la fixation de leurs prix de référence ne prennent pas en compte les prévisions d'évolution quant à la diffusion de ces produits au cours des 3 prochaines années puisque la présent qu'on dément prospective par nature aléatoire nuit en effet, à la limite, lisibilité du dispositif pour les entreprises et pourrait donc nuire à l'attractivité du dispositif attendu qui doit être certes réguler, mais qui est quand même une spécificité française qui permet un accès : un accès à l'innovation pour des patients donc, voilà l'objet de de cet amendement. Merci madame la Ministre votre avis. fait le prix payé pendant la période du prix qui va être négocié après par le CNPF, on s'expose à payer extrêmement cher sont récupérés ensuite sur ce qu'on aura payé pendant la donc ça va exploser, la sécurité sociale, un surcoût considérable et ça risque de mettre en péril le dispositif des athées, je pense qu'il y a un risque, moi je vous propose un retrait sinon défavorable. Madame la rapporteure. au Sénat et et que la commission a accepté de reconduit avec le bureau, je l'espère, bureau du Sénat va bientôt confirmer, nous nous pencherons sur cette c'est problématique datée parce qu'on est sollicité beaucoup aussi par des des laboratoires qui jouent le jeu de l'innovation et qui jouent le jeu de de l'application, par exemple en oncologie pédiatrique du règlement européen, donc nous souhaitons vraiment qu'il y a un travail de fond avec vous, Madame la Ministre, avec Lanka peut-être sur les athées, donc je j'accepte de retirer cet amendement. Merci. Amendement 400. Oui non

pour dire que j'aimerais quand même faire partager Madame une réflexion sur la représentation des usagers au sein du CEP, il semble opportun en effet de mener cette réflexion sur 2 axes de pour 2 raisons principales : d'une part, évidemment, pour renforcer la démocratie sanitaire de la politique économique du médicament, en particulier avec comme objectif d'augmenter la confiance des usagers, ce qui me semble important et d'autre part surtout pour valoriser les innovations à leur juste prix et réduire ainsi le temps d'accès aux marchés innovants et pour éviter toute perte de chance pour les usagers. Très bien, Madame la Ministre. J'ai sports répondra à Monsieur Président Madame rapporteur, bien sûr, nous devons travailler sur la TVA sur les extensions d'indications, il y a urgence est un sujet que nous avons bien identifié et nous serons ravis de partager avec vous, quand nous aurons trouvé une solution, solution, d'autre part sur la représentations des usagers au sein du CNPF je crois que vous avez raison, aujourd'hui, il y a une convention-cadre qui signé entre Monsieur PS : les usagers, on va attendre qu'elle soit signé et nous allons poursuivre à des plus loin, je vous remercie. Très bien donc amendement retiré et maintenant nous passons à l'amendement 400 485 rectifier monsieur Vatrin. Oui, l'article 80 du projet du PLFSS pour 2016 adoptée sous l'ancienne mandature a prévu des temps mais pouvoir conféré aux ARS en leur donnant notamment la possibilité de sanctionner les établissements qui ne s'inscrirait pas dans les contrats dits pour l'amélioration de la qualité de l'efficience des soins ou qu'il le ferait imparfaitement ces contrats conclus entre entraînerait la RS, la Caisse primaire d'assurance maladie, chaque établissement de santé ont pour objet d'améliorer la qualité, la sécurité et la pertinence des soins des prescriptions de permettent la diminution des dépenses de l'assurance maladie, ils comprennent une partie obligatoire relatives au bon usage du médicament une partie composée d'un ou plusieurs volets additionnel, conclu pour une durée maximale de 5 ans, des sanctions sont prévues en cas de refus de l'établissement de coups souscrire ce type de de contrats, par ailleurs, en cas de refus de souscrire un volet relatif aux produits de santé, le directeur général de la RS peut décider de réduire pourcent de leur taux de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, nous considérons que les ARS, créé par la loi HPST dispose déjà de pouvoirs très fort quant à l'organisation de la santé sur le territoire qui n'est pas besoin d'en rajouter, nous contestons la logique de compression des coûts qui prédomine à travers ces mesures et qui s'impose dans la gestion du service public hospitalier que toutes les conséquences que sont constatées peu et par les personnels soignants et par les patients pour ces raisons et en cohérence, d'ailleurs avec notre demande de suppression, l'article 39 que sa collègue Laurence Cohen évoquera dans un instant, nous proposons l'abrogation de cette dispute. Merci l'avis de la commission. en cas de non atteinte des objectifs fixés contractuellement bon les les établissements exemplaires doivent pouvoir recevoir un intéressement, mais il est également utile de pouvoir sanctionner en dernier recours, un établissement qui n'engagerait pas d'évolution de ces pratiques, en effet, ça contribue à la responsabilisation des équipes sur les enjeux de qualité déficiente soins sur lequel il faut faire porter les l'effort dans les, les, les années qui viennent, donc c'est une demande de retrait ou un avis défavorable. Très bien, Madame la Ministre défavorable pour les mêmes raisons, madame la rapporte très bien monsieur mettre : pas de retrait non on vote donc 2 avis défavorables qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, il n'est pas à adopter, nous passons maintenant à la discussion sur l'article 39 avec à nouveau un amendement 480. le groupe communiste. Oui, merci Monsieur le Président, cet article prévoit d'attribuer un intéressement aux établissements de santé qui réaliseront des économies, le montant de l'intéressement sera proportionnelle aux aux économies réalisées, nous savons toutes et tous ici que les établissements de santé sont en en grande difficulté financière. Que le fait de vouloir effectivement que les deniers publics soit bien géré, personne ne peut s'y opposer, mais le problème qui est posé, qui est, qui est devant nous, là, c'est l'offre de soins et la qualité des soins et le fait que les établissements de santé, je pense notamment aux hôpitaux sont littéralement asphyxié alors donner un bon point pour ceux qui font des économies, mais des économies sur quoi pour restreindre quoi si c'est par rapport à la à la la au service rendu et à l'accueil des patients à la qualité des soins, je ne pense pas du tout que ce soit de une bonne, une bonne mesure et vous avez pu le voir durant tout le débat que nous avons depuis lundi sur ce PLFSS 2018, ça n'est pas en tout cas ce qui anime mon mon groupe donc c'est pourquoi dans la logique d'ailleurs que a très bien exprimé Dominique Vatrin, nous ne sommes pas favorables à ce genre de de mesures qui sont contraignantes qui sont inappropriées à la situation des établissements de santé, nous demandons la suppression de cet article.

monsieur le Président, je crois, je rajouterai que si nous supprimons l'article 39, nous arriverons à faire perdurer le régime actuel, dans lequel l'évaluation des cas quesque entreront en vigueur en 2018 reposant uniquement sur des sanctions, donc je pense que ça sera pire encore, de votre point de vue, en tous les cas et donc défavorable. Pas d'explication de vote. Donc 2 avis défavorables qui est pour cet amendement 486. Qui est contre.

Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mis, chers collègues, l'article 39 qui vise à renforcer la pertinence et l'efficience des prescriptions hospitalières s'inscrit dans la continuité de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016, qui avait prévu à son article 81 le regroupement 1er janvier 2018 des différents contrats portant portant sur les produits de santé, les transports et la pertinence et la qualité des soins, on a support contractuel unique, le contrat d'amélioration de la qualité et le et efficience déçoit ce cas 15 qui sera applicable à tous les établissements sanitaires et qui sera conclu entre l'Agence Régionale de Santé l'organisme local d'assurance maladie et les établissements de santé a donc pour principaux objectifs d'améliorer la qualité et la pertinence des soins de simplifier les procédures de contrat actualisation et d'évaluation et de réduire les dépenses d'assurance maladie, le nouvel élan que ce PLFSS entend donner au cas caisse ne doit pas constituer un moyen de pression aux mains des directeurs d'établissements ou des investisseurs, exploitant les établissements privés pour orienter les pratiques selon un unique critère de rentabilité, je m'inscris pleinement dans la démarche d'amélioration de l'efficience et de la qualité des soins, qui vise à optimiser les parcours de soins des patients, c'est pourquoi il ne faut pas que seule une logique de rentabilité soit pris en compte les pratiques les plus rentables ne sont pas nécessairement ni les plus pertinentes, ni les plus efficientes, ni les plus qualitative pour les parcours de soin des patients, l'objet du présent amendement et donc d'exclure de la conclusion d'un contrat toute clause contraire à l'indépendance des praticiens exercent exerçant dans un dans l'établissement de santé. Sans merci,

l'objet d'amendements et que le nouvel élan que la loi de financement pour la suite sociale pour 2018 entend donner au cacao et nous pouvons il y a favorable ne doit pas constituer un moyen de pression aux mains des directeurs d'établissements publics ou des investisseurs, exploitant les établissements privés pour, le cas échéant, vers des pratiques qui ne serait pas médicalement les plus pertinentes, d'où l'amendement, je vous remercie.

la ligne à ligne à l'alinéa 2 le contrat ne contient aucun indicateur qui dépend de la prescription médicale, cet amendement vise donc à exclure les indicateurs liés à la pression médicale de cette liste, merci. Avis de la Commission sur ces 2 amendements identiques, et certains en discussion commune. Ces amendements répondent en effet une préoccupation importante que celle, et verte et de de prescription garantis par le code de déontologie médicale c'est dans cet objectif que je pense à l'Assemblée nationale a été a été prévu que dans le texte soit inscrite et non pas par règlement mais dans le texte, la consultation des commissions et et conférences médicales d'établissement en amont de la signature des caisses parler les établissements de santé, ce qui permet d'associer le corps médical aux objectifs de qualité et pertinence des soins et qui répond à nos yeux, aux interrogations qui sont portés par les auteurs des amendements

l'idée c'est de travailler sur la pertinence et la qualité des soins et pertinent, ça veut dire éventuellement prescrire plus de génériques, ça veut dire s'intéresser à la façon dont un acte et pratiqué éventuellement en surnombre dans un établissement, pourquoi pas, donc l'idée n'est pas du tout de d'empêcher évidemment la libre prescriptions des médecins, la caisse ne déroge pas au code de déontologie médicale mais elle incite les médecins à travailler sur leurs pratiques et notamment sur la pertinence et la qualité des soins, donc nous pensons au contraire que cet outil est très utile pour aller dans le bon sens, en plus, nous avons adopté à l'international, un amendement qui vise à associer en amont, laissez-moi des établissements à la signature du cacao, c'est donc nous avons justement pris soin, le gouvernement était favorable à ce que la communauté médicale soit impliqué dans cette trajectoire dans ce dispositif, et donc, nous vous proposons un retrait parce que nous pensons qu'il n'y a une mauvaise interprétation aujourd'hui de du dans cette dans l'amendement que vous proposez donc retrait défavorable. Madame Damico,

comme vous l'avez dit Divonne Douai peuvent donner un avis préalable à la conclusion d'un contrat, mais il est donc souhaitable que c'est avis ne soit pas uniquement consultatif, comme il l'est en dents en dans le droit mais contraignant.

lui, Monsieur le Président l'amendement est maintenu, nous comprenons bien que les intentions sont louables, quels sont les objectifs que nous pouvons soutenir amendement a pour objectif de prévenir des dérives qui pourraient naître des pratiques suite donc des dispositions qui sont évoquées aujourd'hui. Donc, on passe au vote sur ces 2 amendements identiques qui est pour. Qui est contre On va revoter ce n'est pas très clair, assis, debout, qui est pour.

C'est un autre amendement que je soumets au vote qui est pour. C'était C'était pas les mêmes, nous passons à la discussion de l'article 39. 127 madame de roche. Madame la ministre, votre avis favorable, pas de. Explications de vote qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, il est adopté

Bon, comme. Je l'ai déjà dit la Commission partage bien sûr sur le principe, l'intéressement des établissements de santé avec qualité impertinence des soins, de nature à responsabiliser les équipes sur ces enjeux majeurs toutefois sur la méthode, on a bien vu que la démarche de contractualisation cours à certaines limites et la volonté des ARS, hein, puisque c'était l'objectif fixé de conclure des contrats parfois marche forcée avec l'aide s'établissement avant la fin de l'année pour respecter la date d'entrée en vigueur de ces contrats au 1er janvier 2018 a conduit à une insuffisante individualisation des objectifs, le directeur général de la CNAM l'a d'ailleurs reconnu devant nous des pratiques très hétérogène sont relevés, selon les régions, certaines vont à rebours de l'objectif de simplification et lisibilité des objectifs puisqu'ils ont imposé dans ces cas, caisses d'établissement, le suivi, parfois de plus de 100 indicateurs on aller jusqu'à 150 il serait donc contre-productif en voulant aller trop vite de perd de vue la finalité de la démarche à laquelle, je le répète, nous souscrivons pleinement sur le principe, c'est la raison pour laquelle nous avons demandé le report de l'application des sanctions en cas de non-signature du au 1er janvier 2018 pour laisser le temps à la campagne de contractualisation de se déployer

de ne pas appliquer de sanctions, en 2018, 2019 a été donné aujourd'hui au DG d'ARS lors de leur séminaire par la direction de la déjà et la DSS pardon, donc on est tout à fait pragmatique, l'idée n'est pas de mettre une les les établissements en très grande difficulté et donc je dirais que la mesure sera appliquée avec tact et mesure, donc je vous propose un retrait de cet amendement pour ne pas l'inscrire dans la loi

Qui et contre qui s'abstient, cet article est adopté, nous passons maintenant à la discussion après l'article 39 amendements 296 rectifier bis Monsieur Chassaing. Il est retiré, donc nous passons toujours après l'article 39 au 298 rectifier bis toujours Monsieur Chassaing. Oui, Monsieur le Président, Madame le ministre président cher collègue, la a été institué donc la loi de financement 2015, ce dispositif impose plus de santé indicateurs aux établissements et accentue une pression administrative sur les établissements de santé, donc je propose cet amendement propose donc de repousser l'application des sanctions liées à ce dispositif au 1er janvier 2020. Madame la rapporteure votre avis. Oui, c'était le même que le mien, madame la ministre nous a indiqué, il y a, il y a quelques minutes que que des instructions avaient des données pour que les sanctions soient repoussées instructions données aux ARS, donc c'est une demande de retrait bien évidemment de l'amendement de monsieur Chasse. Madame la Ministre

Oui Monsieur Président : l'application des indicateurs du CAC, c'est très hétérogène, cet amendement propose la création de comités de suivi de l'application de ce dispositif où seront représentés des fédérations hospitalières publiques et privées, merci. L'avis de la commission Madame la rapporteure. Oui, alors on comprend l'objectif d'amendement, mais bon, la création d'même telle comité de suivi nous une doit pas figurer dans la loi ce somme relevait de la bonne gouvernance générale au niveau des du ministère de la Santé, pas le suivi de ce dispositif, c'est donc une demande de retrait. Madame la Ministre votre avis très si voulez favorable pour les mêmes raisons Monsieur Chassaing, vous dites quoi il retire. Donc, article 40. Maintenant, nous passons à la discussion de 2 amendements identiques. Madame Houpert était là, pardon. Pardon, pardon, je n'ai pas encore changer. ça devait m'arriver ça devait m'arriver, chez le président Lana ministre Alain Prost motion du médicament est une activité encadrée par la loi et par une charte de l'information par démarchage protection vivant à la promotion du médicament cette charte est signée par l'État, représenté par le CE, PS et par les industriels, représentés par le cette charte actuellement en vigueur datent d'octobre 2014 la promotion du dispositif médical est une activité également encadrée par la loi et l'article 40 instaure également miroir du médicament, une charte pour mieux encadrer cette activité, l'article 40 prévoit par ailleurs que chaque directeur d'établissement de santé devra définir les conditions de réalisation et d'encadrement de cette activité dans son établissement et que ce processus aura l'obligation de l'objet d'une certification des médicaments et dispositifs médicaux ayant chacun leurs règles leur particularité c'est un amendement vise à clarifier les champs respectif d'application de cette mesure en faisant clairement référence respective ment aux chartes encadrant la promotion du médicament et du dispositif médical. Merci monsieur opère l'avis de la commission Madame la rapporteure. C'est vrai que on a entendu ses réserves sur l'article 40 sur l'encadrement des activités de présentation d'informations.

Et dans la mesure où les discussions relatif en référence à la seule promotion des spécialités pharmaceutiques, il nous a semblé en effet que, qu'on pouvait donner un avis favorable, c'est ça. Bien, madame la ministre, de votre avis. Notre avis est défavorable, la certification par la chaîne des activités de présentation d'informations de promotion en faveur des produits de santé, que ce soit, dispositifs médicaux, médicaments et des prestations qui le rend sont associés à pour but de mieux encadrer les pratiques susceptibles d'inciter à l'achat par les professionnels, donc ainsi qu'il s'agisse d'une présentation ou d'une information, quel que soit le nom qu'on lui donne, il est primordial que cette information soit soumise aux mêmes règles, cela permettra d'éviter tout contournement de la mesure, en effet, on a constaté dans le Champ du médicament que les visiteurs médicaux ont été remplacés aujourd'hui par des médecins de liaison scientifique dont l'activité est en fait très peu encadré sur-le-champ promotionnels, donc nous sommes défavorables à cet amendement. Donc amendement avec l'avis favorable de la commission avis défavorable du gouvernement comme il n'y a personne à pour défendre l'identique suivant nous passons va directement qui est pour Monsieur Savary venu, explications de vote. Oui, monsieur, moi j'ai bien compris l'explication de Madame la Ministre, effectivement, faut être attentif à tout cela mais, a contrario, s'il faut être attentif au décret qui sont pris derrière. J'ai eu l'occasion de voir justement une entreprise chez moi qui fait des dispositifs médicaux et donc aussi des des fauteuils, les fauteuils roulants coquille qui sont maintenant par décret. Qui sont maintenant par décret réservé aux personnes âgées de plus de 65 ans, me semble-t-il et de Geering et de ce qui exclut celles qui sont un petit peu moins dépendante les GIR 4 5 pour 2 personnes j'aime également les personnes handicapées, on voit bien que par le biais de décrets. en tout cas son remboursement à disposition d'autres personnes, donc je demande au gouvernement d'être attentif à tout cela et je souhaite une réponse, Madame la Ministre. Et Madame la Ministre, à vous la parole. Juste pour répondre à Monsieur Savary, vous citez un cas tout à fait particulier, donc ça m'ennuie d'en faire une généralité, mais se trouve que c'est coquille était dangereuse pour la santé et entraîner beaucoup d'effets secondaires, c'est la raison pour laquelle nous avons limité par décret leur usage, donc je vous ai répondu par courrier, vous allez recevoir. Très bien, nous passons au vote donc, monsieur, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, ministre parlait tout à l'heure de pertinence et de qualité des soins, je pense que c'est un amendement rentre tout à fait dans ce cas-là, merci. Donc il est maintenu : avis favorable de la commission avis défavorable du gouvernement qui est pour. qui est pour. Qui s'abstient-il être adopté, nous passons à un amendement de la commission Madame, de Roche, vous avez la parole numéro 130. Oui, là, ça concerne les dispositifs médicaux et nous avons souhaité limiter l'encadrement à la seule activité de promotion de ses produits, puisque la présentation une information adaptée des dispositifs médicaux par leur fabricant constitue déjà une obligation prévue réglementé dans le cadre européen en application notamment de la directive 93 42 du règlement 745, 2017 également de la norme ISO MNEF 14971 Gestion des risques, le risque serait donc alors de créer une double obligation de certificats au contenu identique et je rappelle que les dispositifs médicaux en effet sont très variables en termes de de ce qu'un dispositif médical, on a parlé ces mais ça va, dispositif très innovants, comme les choses toute simple et et beaucoup de petites entreprises sont sur le secteur du dispositif médical, il nous semble que d'avoir cette double certification pouvait alourdir la charge de ces entreprises inutilement. Merci la vie du gouvernement, Madame la Ministre. Oui je je suis défavorable évidemment à cet amendement pour les mêmes raisons que tout à l'heure et je rajouterais en plus que ce qui compte, ce qui est couvert par le règlement européen aujourd'hui sur l'information sur ces produits concernent la sécurité sanitaire et pas du tout l'usage, la pratique ou la pertinence de cet usage et donc le règlement européen ne couvre absolument pas le Champ aujourd'hui couverts par achat donc toujours défavorable à cet amendement.

Qui est contre qui s'abstient l'amendement était adopté, nous allons finir la matinée avec une discussion commune de 4 amendements dont trois identique, la parole est à.

qui prévoit qu'au regard notamment de l'intérêt de la santé publique de l'impact financier ou des risques de Meuse Hysaj la prise en charge d'un produit de santé de ses prestations, éventuellement associés puisse être subordonnée au renseignement par le professionnel de santé sur l'ordonnance d'éléments relatifs au contexte soit la motivation de la prescription, ces éléments présents sur l'ordonnance doivent être transmis au service de du contrôle médical par le prescripteur, le pharmacien ou le cas échéant par un autre professionnel de santé, selon une forme qui sera déterminé par voie réglementaire, par ailleurs, cette obligation est assorti de sanctions en cas de non-respect, il nous apparaît que cette disposition est extrêmement chronophage pour les médecins et les professionnels de santé concernés et qu'elle constitue une charge administrative considérable au détriment du temps consacré aux soins par ailleurs en obligeant le médecin a motivé le pourquoi du comment de sa prescription, elle tend à remettre en cause à la fois la liberté de prescription, mais aussi le secret médical. amendement 233 Monsieur Morisset. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre je j'ai pas reprendre ce qu'a dit notre collègue sur le pourquoi de cette amendement veut simplement reprendre le texte, elle qui nous est proposé aux lanières 31, il est dit que la prise en charge par l'assurance maladie peut être sur Bordeaux, il y a pas d'obligation, il peut être subordonnée mais après on dit qu'il est subordonné, pourquoi professionnel de santé détecte qu'il aurait un impact financier alors c'est quoi un impact financier pour le professionnel de santé et surtout à l'année à 33, il a dit que si le non respect de ses obligations, peut donner lieu à un constat d'abus, j'arrive pas à comprendre que, dans un article, on m'aider peut un peu partout et puis qu'à la fin, on parle de sanctions s'il avait doit je suis d'accord doit être subordonnée mais c'est peut-être subordonné, je vois pas comment les professionnels de santé pourront effectivement apprécier dès lors qu'ils doivent le faire quand il y aura un impact financier et puis, surtout, le professionnel de santé doit expliquer ensuite apporter une raison pour laquelle il prescrit cette ce médicament donc voila pour quelle raison cet amendement, je soutiens sans problème. Madame Delmont-Koropoulis pour un amendement identique.

Oui, alors le il est en partie rédactionnelle parce qu'il vise, en outre, a précisé les conditions relatives à la constitution de l'obligation de renseignements de l'ordonnance pour la prise en charge des produits prescrits. ça rejoint, ça rejoint un peu les les amendements précédent mais en précisant le Vous dites donc que vous donnez un avis favorable aux trois identique précédent. Lancé un avis de sagesse corps vie favorable au miens. Oui, ça, madame la ministre, votre avis sur l'ensemble. Mon avis est défavorable, mais je souhaite expliquer l'esprit avec lequel cette mesure a été faite, nous avons plusieurs sujets, nous avons aujourd'hui des médicaments qui peuvent être prescrits en ville et qui sont horriblement coûteux pour l'assurance maladie, je pense à certains anticorps monoclonaux dans la semaine par exemple dans les instances, dont l'indication excessivement restreint, et nous n'avons aujourd'hui aucun moyen de contrôler ces médicaments, donc cela permettrait d'endettement, cas exceptionnel de demander aux médecins de stipuler l'indication de ce sera donc une une demande du ministère, ça n'est pas du tout une mesure qui vise à mettent les indications pour l'ensemble des ordonnances, bien entendu ça sera informatisé, ce sera un dispositif d'exception et la raison, pour lequel je suis défavorable à l'amendement même de recherche, en fait, nous avons un 2ème souci en dehors des médicaments extrêmement coûteuse c'est le mésusage et notamment le mésusage des antibiotiques, aujourd'hui, nous savons que les prescriptions sont trop longues, que, il y a prescription d'antibiotiques à très large spectre pour des indications qui ne sont pas les bonnes, et donc nous avons besoin d'avoir une vision et un meilleur contrôle de l'usage des antibiotiques en ville, notamment pour les affections courantes et donc c'est vraiment un dispositif qui vise à régler, soit des problèmes liés à l'impact financier de certaines prescriptions soient à l'impact de santé publique, alors il n'y a pas de questions sur le secret médical totalement couvert par l'ordonnance puisque l'ordonnance élu par un pharmacien qui est couvert évidemment par le secret médical, ce sera très simple puisque le nouveau référentiel des logiciels d'aide à la prescription permettra en fait d'intégrer l'indication dans les ordonnances que lorsque ce sera demandée

Oui, compte tenu de ce qui vient d'être dit sur le sujet, peut-être, mais je Cannes pavé dans la mare, mais faudrait-il s'interroger un jour soit la sacro-sainte liberté de prescription. Bien, alors je veux quand même donner une précision à Madame. Je veux Je veux donner une précision, c'est que vous avez donné un avis de sagesse. Si ces amendements identiques passe le votre tombe, on est d'accord.

majeur que celui du mésusage, donc moi je vais retirer l'amendement combien ça pèse 196 c'est ça parce que j'ai bien compris, néanmoins, il faut reconnaître, Madame la Ministre, que la formulation de l'article telle qu'il est défini, ce que vous dites et pas si évident que ça pour les professionnels de santé et il y a des craintes qui ont été fortement exprimée sur cet article 40 à la fois par les les professionnels enfin les, les producteurs, dispositifs médicaux mais aussi par les professionnels de santé et par notamment si tout ce qui tourne autour de de 10 de de soins de missiles et autres, donc ça on comprend quand vous l'expliquer ce que vous dites quand on lit l'article n'est pas forcément suivez donc ça, néanmoins je vous fais confiance à vous professeur de médecine, je retire mon amendement. Mais si si vous retirez le vôtre, vous maintenez la sagesse sur les autres avant qui disait la même chose à peu près, j'aimerais savoir.

Vous avez bien vu, monsieur le président, chaque que le positionnement de de la rapporterait est un peu compliqué par rapport au texte écrit et par rapport à à l'explication de texte donné pas madame la ministre, en fait, il y a la personnalité juridique du texte qui n'est pas fait mais qui et l'explication médicale de la professeur de médecine, qui était donné ensuite : on veut bien se ranger au côté médical, explication qui est donnée par Madame Buzyn en en disant quand même que le texte de la ministre et le moins, on a moins confiance autre examiner ce qui est l'explication d'un professeur.

la commission demande le retrait de ces amendements identiques à retirer celui qu'elle avait déposé, le gouvernement est défavorable à ces trois identique Alesi Monsieur Morisset. Attendu d'explication de Madame la ministre, et moi je, je, je maintiens mon amendement pour quelle raison, parce que même si vous faites une liste par voie réglementaire et dédié à l'article 1er que la prise en charge, peut-être alors toute façon j'arrive pas à comprendre, il faut au moins mettent le mot devra, dans la mesure où vous arrêterez par voie réglementaire, une liste de médicaments, c'est pour ça que je maintiens mon amendement pour y voir clair dans la formulation juridique ensuite qui pourra intervenir à une autre occasion rassurer un petit peu nos professionnels de santé pas mettre un article avec 3 alinéa pour mettre peut-être. Donc, donc les autres amendements identiques sont maintenus. Oui, monsieur le président, moi je souhaite que la médecine soient réservées aux médecins et même pas voter avec des des cadres au aussi contraignant. Bon, très bien, de toute façon, on passe au vote qui est pour ces amendements identiques. Qui est contre. Qui s'abstient ils sentent. Je vais suspend la séance, elle sera reprise à 14 heures 30 pour la suite de l'examen de ce texte, la séance est suspendue.